L'ordre du jour appelle l'examen des demandes de la Commission de la culture de l'éducation et de la communication et de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat en application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 58 relatives au fonctionnement des assemblées parlementaires qui leur confère pour une durée de 6 mois les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener une mission conjointe de contrôle afin d'examiner la question du signalement et du traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes. Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de la séance du 14 juin dernier. Je vais mettre aux voix. Les demandes de la Commission de la culture de l'éducation, de la communication et celle de la commission des lois qui est pour. Qui est contre. Elles sont adoptés en conséquence la commission de la culture de l'éducation et de la communication et la commission des Lois se voit conférer pour une durée de 6 mois les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener cette mission conjointe de contrôle le gouvernement sera informé de la décision qui vient d'être prise par le Sénat. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à assurer la pérennité des établissements de spectacle cinématographique et l'accès au cinéma dans les outre-mer présenté par Madame, Catherine Conconne et plusieurs de ses collègues demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Dans la discussion générale. La parole est à Madame, Catherine Conconne, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre délégué. Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs, chers collègues. Permettez-moi avant tout de remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis à cette initiative de prospérer. Qu'il s'agisse de mon groupe politique, qui m'a ainsi volontairement. Cette priorité dans la niche du jour mais aussi des différents ministères et des différents professionnels auditionnés. C'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui cette proposition de loi. Un en car. Suzanna bon qui pourrait paraître technique. Ce texte est en réalité très symbolique pour ce que l'on a l'habitude d'appeler les outre-mer. Le texte que je porte devant vous, parle de culture dans des territoires où l'offre culturelle est plus réduite et où elle repose sur des acteurs fragiles qui se battent pour la faire vivre au quotidien. Pourtant, vous le savez, la culture est nécessaire à l'être humain. Le père de la nation martiniquaise disait qu'est-ce que la culture, hé bien la culture à la vie vivable et la mort. Ah frontales. Elle repousse les horizons ouvrent les imaginaires. Elle doit à ce titre et dès que nécessaire. Être préservé des règles qui régissent l'économie la France le sait bien, n'est-ce pas Monsieur le Ministre. Elle qui est à l'origine du concept d'exception culturelle. Ce principe qui fait de la culture bien à part qui ne peut être soumis au fonctionnement classique du marché. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La préservation de l'accès à la culture dans les Outre-mer. Je vous parlerai aussi de Vichères dans nos territoires, le coût de la vie est telle que de nombreuses familles consacrent l'intégralité de leurs revenu aux seules dépenses dites essentielles, logement, nourriture, transport et parfois cet accord est suffisant pour couvrir les besoins. Alors autant vous dire que les dépenses culturelles sont loin souvent d'être prioritaire. Malgré tout le cinéma reste loisir relativement accessible et constitue une sortie prisée des familles des jeunes ou des scolaires. Les cinémas vont monter dit trois ans sont devenus des lieux de vie dynamique qui développe des activités et crée des événements et rassemble des publics extrêmement divers. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui assurer leur survie voilà plus d'un an que les cinémas des Outre-mer doivent affronter une attaque commerciale coordonnée de la part des principaux distributeurs notamment américains dans les films représentent la majorité des entrées en salles chez nous ces multinationales puissantes ont entrepris d'augmenter brutalement le taux de location que les cinémas leur reverse et qui correspondent à une part des entrées réalisées pour chaque film cette pas été fixée chez nous a historiquement 35% un niveau qui permet à la fois aux distributeurs de rémunérer légitimement aux exploitants de salles de se développer tout en maintenant un prix des tickets abordable sans aucune contrainte légale et sans des acteurs concernés ce taux s'est naturellement imposé sur tous les territoires, car il correspond à une réalité économique, aujourd'hui les distributeurs souhaitent l'augmenter de 15 points pour le faire passer à 50% au cours des premières semaines de diffusion des films comme cela se pratique dans l'Hexagone. Une telle augmentation qui n'est justifiée par aucune urgence ni aucune nécessité économique, serait évidemment inabsorbable par les exploitants de salles. C'est d'autant plus vrai qu'elle intervient suite à la crise du Covid, qui a conduit pendant 2 ans. Oui, 2 ans, à une désertion des salles de cinéma avec des taux de fréquentation au plus bas chez nous cette réalité est d'autant plus marquée que dans l'Hexagone et ça peine encore à retrouver leur public d'avant crise. Dans ce contexte, une augmentation des taux conduirait à la fermeture rapide de plusieurs établissements en Guyane. Mon cher Georges. En Guadeloupe, les 100 des Thierry trois son cinéma in augmentation conduirait à l'arrêt des projets d'investissement porté par ses exploitants et à un rétrécissement encore de l'offre culturelle proposer à nos populations en 2018 un rapport de la très respectable expression générale des finances avait d'ailleurs mis en avant la faible rentabilité des salles de cinéma ultramarines et préconisait déjà oui 2018 un taux plafonné de location nos établissements de cinéma ont tenté de négocier pendant plusieurs mois en lien avec le CNC pour trouver un compromis et éviter le pire, mais les distributeurs n'ont rien voulu savoir et le pire est devant nous dans les négociations. Ils sont en position de force. Grande Marjan internationale face à des petits exploitants locaux la discussion est inégal. Les distributeurs peuvent imposer les 50%. La bataille est perdue d'avance. Le pot de terre s'affrontent au pot de fer. Quand le marché ne permet pas de trouver une solution satisfaisante en matière culturelle. C'est à la puissance publique d'intervenir. L'État ne peut abandonner sur le bord de la route des marchés fragiles à l'autorégulation. La force de la France. Monsieur le Ministre, se trouve dans cette culture de la protection de la solidarité et d'une recherche permanente et légitime des cette notion d'équité a du sens pour nos populations. Je ne viendrai pas ici vous rappeler nos existences qui porte encore des stigmates Frath frappée d'injustice lors de la grande crise sociale de 2009 un néologisme légitime était née du sentiment de révolte d'une résignation étouffante. On avait parlé de profitation. Alors à tout moment dans tous les domaines, les enfants de ces pays qui se trouve en responsabilité et je me sens concerné doivent s'assigner la tâche de traquer en permanence tout ce qui pourrait contribuer à cette impression légitime. Permettez-moi, à ce titre de merci votre action. Monsieur le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco. Hier, nous nous battions pour une continuité territoriale mieux assumée par l'État pour assurer les déplacements coûteux de nos compatriotes sur les territoires des initiatives sont prises et vous vous impliquez énormément dans cette dynamique pour réguler les éléments de Vichères, tous acteurs confondus avec par exemple le bouclier qualité/prix appeler chez nous. Bé Cuper. Il nous faut poursuivre oser être audacieux bousculées, parfois l'ordre établi. Chez nous on dirait Maroni. Nous ne pouvons assister résigné à la disparition de nos salles de cinéma, notre loi est une loi légitime notre loi est une loi de bon sens. Elle vise à plafonner les taux de location en mer à leur niveau historique de 35% et à assurer la pérennité de nos établissements. J'entends ici et là des décrète avec notre texte. Les distributeurs ne pourraient plus on ne voudrait plus distribuer leurs films dans les outre-mer moi je leur dis, il n'y aura pas de chantage sur ce sujet. Quel argument étonnant c'est le taux déjà en vigueur depuis des décennies les distributeurs le pratiquent déjà. Et si il refuserait tout à coup, ce qu'ils acceptent depuis si longtemps et pense qu'on l'aurait pose de renoncer à quelques gains supplémentaires à une profitation supplémentaires il priverait donc nos populations d'Outre-Mer de l'accès à leurs films. Je n'ose envisager ce scénario et préfère croire qu'une fois ce tumulte passé chaque retrouvera le chemin de la raison saura rester en effet raisonnables et que nous pouvons tous nous retrouver sur la même volonté d'élargir l'accès au cinéma dans le territoire, nous en sortirons tous gagnants et j'insiste grandit exploitant distributeur et citoyens. Je me félicite que ce texte est convaincu en commission et je me permet à ce stade de remercier l'implication sans faille de ma collègue éprise de culture, chef de file pour mon groupe. Sylvie Robert, j'espère que le Sénat qui a aussi accordé un avis favorable très large en commission sera aussi partager nos objectifs nos territoires dits d'outre-mer nous regardent, ils attendent qu'on sache les protégés, ils attendent qu'on les défende là. Culture aussi chez nous. Ne les décevrons pas. Merci. Bien me monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi de notre collègue Catherine Conconne, je la remercie vraiment vraiment de l'avoir déposé car en réalité, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous n'aurions peut-être pas dû examiner cette proposition de loi, vous l'avez compris, elle approuve objet de préserver les conditions via pour l'exploitation cinématographique dans les outre-mer mais elle est surtout en réalité la conséquence de l'échec des négociations menées cet Automne sous l'égide du CNC entre des acteurs pourtant habitué à collaborer et à travailler ensemble pour faire vivre le cinéma, je parle bien sûr des exploitants et les distributeurs.

Rapport qui met en valeur le rôle pourtant central mais encore mal connue des distributeurs. Ces derniers constituent en effet le chaînon entre la production d'un film et son accès aux salles ils occupent des fonctions cruciales qui les mettent en contact avec l'église exploitants et les producteurs. La rémunération des distributeurs repose sur une fraction du prix du billet dans une fourchette fixée par la loi entre 25% et 50%. Elle leur permet également de faire remonter les recettes vers les producteurs. En métropole, la fraction qui leur revient varie en fonction des films et de la semaine du sortie pour s'établir en moyenne autour de 47 pour 153% revient donc aux exploitants toujours en moyenne. L'outre-mer se singularise pour des raisons historiques que j'ai développée dans mon rapport de 2 manières. D'une part la fiscalité est moins élevé avec un taux de TVA de 2,1% contre 5,5% en métropole et une taxe sur les billets perçus par le CNC de 5% contre 10 72 % en métropole en métropole comme le prix du billet est plus élevé en outre-mer il en résulte une assiette plus avantageuses à se répartir entre les distributeurs et les exploitants. D'autre part, là encore pour des raisons historiques, la distribution a longtemps été assumé au niveau local souvent par les exploitants eux- mêmes qui supportaient donc les frais de promotion dès lors au lieu d'un taux moyen en Métropole de 47% celui en vigueur en outre-mer s'est établi effectivement à 35%. Répartis à parité entre le distributeur national et le distributeur local, en accord avec les exploitants. Il faut le souligner, un terme a cependant été mis à ce système spécifique et les distributeurs ont souhaité assumer directement les actions de promotion des Oeuvres dans les départements d'outre-mer. C'est dans ce cadre que des négociations ont été menées afin de définir les nouvelles relations entre les exploitants et locaux les distributeurs avec pour thème principal, la répartition des recettes issues de la salle. C'est ici le moment de rappeler un fait bien connu de notre assemblée et auquel nous avons toujours comme représentant des élus locaux accorder la plus grande attention. Je veux parler des conditions spécifiques du développement économique en outre-mer notre collègue lady marcher trois contraint de construction de sécurité niveau des salaires, la vie est chère en outre-mer et l'activité économique en tort trop difficile. Dans le cas des cinémas. Cela se traduit par des coûts d'exploitation plus élevés. Plusieurs rapports des inspections générales de l'administration et des finances ont soulevé ce point hé bien montré en tout état de cause que l'exploitation en outre-mer était plus onéreuse. Dès lors, les négociations engagées devait tenir compte de 2 paramètres. D'une part la volonté bien naturel des distributeurs d'améliorer leurs revenus tirés de l'outre-mer en contrepartie il faut le rappeler d'investissement qu'ils devront dorénavant consacrés directement à ces territoires. Mais d'autre part la nécessité littéralement vital pour les cinémas d'outre-mer de poursuivent une exploitation économiquement viable. En dépit je crois pouvoir l'affirmer de la volonté de chaque partie de parvenir à un accord, la négociation a échoué. Les distributeurs ont souhaité pouvoir bénéficier d'un retour plus important ainsi que de marge de négociation que rend difficile un taux de 35% de leur côté une très large majorité des exploitants, a fait valoir le risque je crois avéré de très forte déstabilisation de de l'exploitation cinématographique en outre-mer avec un taux aligné sur la métropole. Comme je vous le disais monsieur ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi et donc une réponse à une situation bloquée où il nous est demandé, en tant que législateur de prendre position. Nous pouvons le regretter car dans cette affaire. Un accord aurait dû. Peut-être devrait encore je suis optimiste, vous le savez, pouvoir être conclu. Je rappelle en effet le développement de la salle est un enjeu majeur singulièrement dans ces départements qui ont un accès moins aisé à la culture. Je regrette d'avoir assisté comme certains d'entre vous à une scission entre les distributeurs et des exploitants, qui devrait être des partenaires mais également entre des exploitants puisque au moins l'un d'entre eux n'a pas souhaité se joindre à la demande. Je tiens cependant à relativiser, pour les distributeurs, les conséquences de cette proposition de loi d'un côté les départements concernés ne représentent que 1,7% des entrées au niveau national. De l'autre côté, compte tenu du différentiel de fiscalité. Je vous en ai parlé et un prix de billet plus Elbé la part qui revient aux distributeurs en outre-mer avec un taux de 35% seraient quasi identique à ce qu'il perçoit en métropole avec un taux de 47%. De cet euro. Contre de. 70 euros. Cela constitue donc pour les distributeurs. Une amélioration nette par rapport à une situation où il ne touchait que la moitié des 35%. Alors il ne faut pas sous-estimer le risque pourrait peser sur l'exploitation en notre mère. Les distributeurs pour en effet choisir de moins s'impliquer dans le cinéma, avoir de moins distribuer. Ce risque existe, il ne faut pas le nier. Nous en sommes conscients et les exploitants premier. Cela dit, je note en dépit de ce risque qu'une écrasante majorité souhaite prendre le chemin tracé par cette proposition de loi, ce qui en dit long je crois sur cette menace existentielle qui pèserait sur alors, mes chers collègues. Au nom de toutes ses valeurs et ses principes qui sont absolument essentiels dans notre assemblée. Je vous invite à soutenir cette proposition de loi qui s'avère nécessaire pour préserver les droits culturels en outre- mer je vous remercie. Merci madame la rapporteure. La parole est maintenant à Monsieur le Ministre, Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer. D'abord peut-être une bonne nouvelle, c'est l'adoption. Conforme à la proposition de loi, madame la présidente Gatel tout à l'heure à l'Assemblée nationale où j'étais où j'ai obtenu la suppression de tout. Le désir d'amendements au nom de l'efficacité législative. J'espère que si cette. Proposition de loi est adopté, ce matin il en sera de même lorsqu'qu'elle aboutira au à l'Assemblée nationale. Monsieur le président. Je suis président de la commission des lois. Monsieur le président de la commission culture madame la rapporteure. Chers Catherine Conconne. Le cinéma, c'est l'heure de sculpter le temps. Écrivit un jour Andrej Tarkovski un des plus grands réalisateurs universel. Depuis mon 1er jour à ce ministère. Je m'efforce en plein accord avec les parlementaires. Avec la ministre de la culture avec les associations, les artistes, les élus locaux, les forces vives de ces sociétés ultramarines. Si enrichissante. Si attrayante de faire du levier culturel, un des moteurs centraux de l'action publique du gouvernement outre-mer. Parmi les mon ministère soutient le cinéma représente un cas particulier, c'est un des derniers venus. Dans la panoplie des arts que le concours des siècles a su dresser pour la contemplation des générations. Il ne date que d'un siècle. Mais avec quel panache a-t-il et qu'il rentré dans l'imaginaire de nos compatriotes de toutes générations, de toutes origines, de toute aspiration. Il est rentré avec son cortège surtout de dizaines de métiers manuels intellectuelles artistique artisanaux. Il s'y est engouffrée avec le désir de peindre la vie comme de la changer d'inspirer les rêves comme de les réaliser de transfigurer la réalité comme de la condamner. Le cinéma est un art total. Peintures et sculptures poésie et musique. Et il ne servirait de rien de continuer à agir pour nos territoires ultramarins. Si tout n'était pas fait pour que le 7ème art qui installe comme chez lui. Le cinéma est un art. Mais c'est aussi une industrie, rappelons-le. Génératrices d'emplois les négociations commerciales. Le partage de valeur ajoutée de rapport de force et je me plais à souligner l'engagement de France 2030 sur des studios de création qui vont se répartir outre-mer. Bref la régulation publique doit donc être assuré partout sur le territoire français, même le plus éloigné d'ici. Comment. Quand à ton accès à Oeuvres d'Simone cinématographique dans nos territoires ultramarins. Cette question doit guider notre action dans la place que le cinéma qui depuis peu dans la vie de nos compatriotes et désormais important. On se résigne trop pas penser qu'une forme d'art arrivera de toute façon dans nos territoires ultramarins. Avec le temps avec de la chance avec quelques incitations avec le hasard des conjonctures. Qui trop souvent et nos audace. Mais parfois il est temps de Suisse. Pendant la chance d'actionner la volonté, c'est la proposition de loi de Catherine Conconne. Le cinéma, c'est l'art de recul sculpté le temps hé bien les populations ultramarines. Aimerait continuer à l'éprouver chez eux. C'est pour réaliser cette mission que la commission culture, de l'éducation, de la communication de votre haute assemblée a adopté le 7 juin 2023. La proposition de loi qui vous est présenté aujourd'hui. Visant à assurer la pérennité des établissements cinématographiques et l'accès au cinéma dans les outre-mer des collectivités concernées sont celles mentionnées à l'article 73 de la Constitution. Il devrait dans le monde idéal de l'économie de l'industrie culturelle exister une liberté. Commerciale par une liberté des prix dont résulterait une juste rétribution des recettes d'un film en le producteur distributeur et exploitant. Le code du cinéma et de l'image animée. En ses articles 213 9 213 à 213 13. Encadre toutefois cette liberté. La taxe sur la valeur ajoutée réduite, avec un taux de 5,5%. S'y ajoute la taxe sur les prix des entrées aux séances la fameuse taxe spéciale additionnelle TSA taxe affectée au fonds de soutien au CNC et de l'image animée, qui se monte à 10,72%.

C'est alors seulement que l'exploitant distributeur bien se mettent d'accord pour définir un taux de location que l'exploitant accordera aux distributeurs négocier l'article L 213 11 du code du cinéma d'iPod dispose que le taux de la participation proportionnelle et librement débattu avec un minimum de 25% et un maximum de 50%. Tout le débat aujourd'hui porte sur la portée de ce librement. On fait beaucoup. État de la liberté dans notre société c'est tant mieux. Ce mot porté depuis 1789 avec talent par nos pères fondateurs. Éric toute la société doit fonder nos efforts et nos projets mais nous n'aurions plus ni utilité ni estime. Si nous dussions échoué à identifier la liberté tant désiré. Face à la licence de dominer de celui qui utilise trop une position avantageuse et pousse trop loin un bénéfice ou un intérêt. Je souhaite partager avec vous l'idée et le fait que l'action publique entre en scène lorsqu'elle a un doute sur l'équilibre des échanges et la justesse d'un accord obtenu ou bien si l'intérêt général le requièrent ou bien si les lésés. Il me semble que c'est le cas ici.

Cette différence ancienne et justifiée par les nombreuses spécificités ultramarines. Non. Dans le cinéma comme ailleurs on ne parvient pas à faire vivre nos compatriotes ultramarins avec les règles de tout le monde. On s'y efforce bien sûr mais on n'y arrive pas toujours. Nous sommes ici pour savoir s'y résoudre et le faire quand c'est nécessaire. 21 établissements seulement 1% du parc national, 1,7% des entrées au cinéma, mais derrière ces chiffres se cachent l'infinies des imaginaires et des des expressions Sensible que nous ne saurions mutilé. la sécurité. La sécurité les charges exploitation du bâtiment par exemple. L'usure du matériel accélérer le surcoût d'investissement. Anticyclonique parasismiques. Ainsi des éléments liés à l'éloignement, le délai des pièces détachées la nécessité de groupes électrogènes fort coûteux toutes ces charges supplémentaires auraient mis en péril depuis longtemps. Tous ces équipements culturels. Si la République n'avait pas réagi en adaptant certains dispositifs. TVA à 2 virgule au lieu de 5,5 et taxe sur les billets calculé de manière différente. L'article 200 de la loi de finances pour 2019 établit ainsi le montant de la TSA à 5%. Cette différenciation du modèle économique. A été objectiver dans un rapport de 2018, commandée par le CNC qui recommandait déjà qui ont commandé déjà en 2018 le plafonnement dans la loi du taux de location des films. Le rapport, précisé que, malgré ces différenciations les salles de cinéma ultramarines, avec une faible rentabilité par rapport aux salles de l'Hexagone. Il préconisait déjà. Déjà. Un plafonnement des taux de location dans les départements et régions d'outre-mer ce rapport constitue un effort d'objectivation. Et c'est celui-là que nous ne pouvons pas ignorer. La présente, proposition de loi propose ainsi, et j'en remercie madame la sénatrice Catherine Conconne. Un régime spécifique pour les exploitants dans les mer, c'est-à-dire un taux de location qui au lieu d'avoir la faculté de monter au gré des négociations jusqu'à 50% serait plafonné à 35%. Ces chiffres n'ont pas été choisie au hasard. Le dialogue avec tous les acteurs de l'industrie cinématographique a duré des années. En ce qui me concerne, depuis que j'ai pris mes fonctions, les parlementaires le savent. J'ai essayé d'accorder les positions de comprendre les manques d'imaginer les possibilités. La solution proposée par ce texte me semble sage. Le CNC engagée depuis l'été 21. Un dialoguant avec l'ensemble des partis aux côtés de la médiatrice du cinéma. Et les différents acteurs, le contexte était complexe. Mais. Nous ne sommes pas venus pas parvenus à un accord, comme vous l'avez souligné madame la rapporteure. Même si les positions se sont rapprochées. Aujourd'hui tout le monde est d'accord pour réfléchir. À l'évolution du modèle de la sous-distribution par exemple. Mais il nous faut avancer maintenant. Cette mesure n'épuisera bien sûr aucunement la marge de négociation du distributeur et exploitant plusieurs outils existent dans la liberté commerciale jours ou semaines de décalage sorties contraintes diverses de distribution montant forfaitaire minimum avec le sous-, distributeur. La discussion ne sera pas bloqué. C'est ce que je veux dire fortement par l'adoption de ce texte. La discussion au compte. Frère pourra continuer plus utilement. Mais aujourd'hui les risques de fragilisation des exploitants sont réels. Et c'est plus que de la fragilisation, c'est un danger de mort. Et ils sont bien documentés dans les éléments que nous avons tous sur des skis les cinémas ont subi des restrictions plus longue que certains territoires situations sanitaires plus difficiles touchant la fréquentation cinématographique et donc les recettes directes qui sont en baisse même si ça remonte un petit peu ces derniers mois. Il nous faut nous en féliciter. Nous sommes un taux de fréquentation proche de celui d'avant crise. Mais il nous faut quand même avancer et avancer. Tout le monde a de métier, le sien, celui de critique de cinéma hein cria a écrit un jour le sénateur, le réalisateur, C'est dire si le cinéma n'est pas un art comme un autre. Il ne transforme pas le spectateur en sujet passif mais en conscience active toujours prompt à sortir de la salle en esprit désirant partager comprendre disséquer ce qu'il a vu et entendu. Privés nos compatriotes. Ultramarins de l'enrichissement de leur imaginaire ne serait pas qu'une paresse. Mais ce serait une grande erreur. Trouver un équilibre entre les acteurs de l'industrie du cinéma n'est pas chose aisée. Et peut être. Et qu'il trouvait grâce à vous, je le pense et je vous en remercie. Après mon aventure à l'Assemblée nationale ce matin. Je suis obligé de partir à La Haye défendre encore une fois les territoires ultramarins avec nos amis néerlandais. Et donc je pense que le ministre il Hechter nous l'attendons me suis plaira dans la. L'exposé des. Raisons de votre de chacune des des groupes de ce cette assemblée merci. Merci monsieur le ministre et bon vent à la. Dans la suite de la discussion générale. La parole est à Madame. Sylvie Robert pour le groupe socialiste pour six minutes. Bien monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'interviens maintenant en tant que chef de file de mon groupe. Vous savez, je suis toujours ravi quand on parle de culture dans cet hémicycle ce moment c'est plutôt souvent donc ça me ça me ravit et encore plus parler d'outre-mer et cette proposition de loi à l'immense mérite d'allier les 2 à la fois de parler de culture et de cinéma donc en outre-mer j'aurais préféré que ce soit une autre occasion parce que cette PPL effectivement une dernière chance de sauvegarder l'exploitation cinématographique en août mais en outre-mer je ne vais pas revenir sur ce que j'ai développé en tant que rapporteur tout à l'heure mais la situation est périlleuse dans un contexte de reprise post-Covid. Au fond, quel est l'objet de cette proposition de loi de préserver l'exploitation cinématographique ultramarines me répondrez-vous mais par delà quelle finalité légitimerait une intervention du législateur dans la relation entre le distributeur et l'exploitant. l'accessibilité des populations ultramarines au cinéma et partant à un des piliers de la culture et de l'art français. Certains aiment à penser que le législateur affectionnent de se mêler de tout. À titre personnel, je crois surtout qu'il a qu'il doit intervenir par nécessité et qui le conduit l'État à assumer le rôle essentiel qui est le sien aujourd'hui celui de régulateur. On le voit sur la question numérique. On est en train d'y travailler, hé bien il en va de même de l'exploitation cinématographique en outre-mer nous devons intervenir par nécessité. En effet, sans cette PPL il est une certitude, la plupart des exploitants ultramarins peut être même tous ne survivrait pas ne survivront pas un relèvement du taux de location autour de 50% à moins d'augmenter le prix du billet à un niveau tel que le public ne sera pas au rendez-vous. Or sans exploitant pas de salle de cinéma. Pas de diffusion. Pas de public et donc pas de culture. Pouvons-nous prendre ce risque et prend le parti du lycée faire en tant que garant de l'intérêt général qui naît en l'espèce, ni celui Denis distributeur ni les exploitants mais bien celui des populations ultramarines, qui ont le droit comme les métropolitains d'accéder au 7ème Art et de voir les films qu'ils désirent. Ma réponse, mais qui est également monsieur le Président, celle de la commission culture est clair et sans ambiguïté, nous ne le pouvons pas et nous ne le devons pas. Comme souligné l'IGAD dans un rapport de 2013 sur l'extension aux départements d'outre-mer des dispositifs de soutien au cinéma du CNC. Je cite l'offre cinématographique est limitée et contrainte dans son développement, alors même que la sortie au cinéma semble être une tradition culturelle forte, forte, laquelle a d'ailleurs entraîné l'implantation de nombreux points de projection fixes ou itinérants au cours des années 50 et des années 60. Aujourd'hui ce passé cinématographique est particulièrement mise à mal alors qu'en métropole, la densité d'équipements moyenne et d'un écran pour 11.340 habitants. Elle n'est que d'un écran pour 27.300 habitants en outre-mer et en plus il y a des disparités. Vous savez très forte en les entre les différents territoires ultramarins. À cette situation s'ajoute les surcoûts structurels, liés au Tom on en a parlé insularité 3 étroitesse des marchés normes antisismiques anticyclonique, coût élevé de la vie en outre-mer rendre accessible la culture et donc d'abord un enjeu matériel très concrets qui concernent l'ensemble des champs artistiques et moi qui suis très attaché aux bibliothèques et aux livres, vous le savez, le prix du livre notamment est nécessairement plus élevé en métropole du fait du coût du transport en ce sens un débat en séance publique sur l'accessibilité culturelle en outre-mer comme Rennes par la commission de la culture à la délégation outre-mer serait pertinent afin d'établir un état des lieux de lever les freins existants et de réfléchir peut-être à la création vraiment de dispositif de compensation qui favoriserait la diffusion de la culture dans ces territoires. Vous l'aurez compris à travers le plafonnement du taux de location qui est proposé dans cette PPL mesure a priori technique nous tendons vers l'idéal politique inscrit à l'ennemi a 13 du préambule de la Constitution de 46, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture et si nous, législateurs ne me donc passer de bataille qui la mènera néanmoins j'entends les appels à la vigilance quant aux répercussions de cette PPL sur la diversité culturelle singulièrement sur la diffusion des films indépendants. C'est ce que nous a dit j'y suis sensible mais comme en métropole. Le public ultramarins doit avoir un large choix entre les blogbuster, on en a parlé. Les films populaires mais aussi les films d'auteur, il est hors de question de renoncer à cette diversité et nous devrons peut être évalué l'impact de cette PPL en la matière. J'ajouterai enfin que la prise en considération de la diversité culturelle doit être réciproque. Et là je m'explique. Si les films d'auteur d'origine métropolitaine ont vocation à être diffusée en outre-mer les films ultramarins ont tout autant vocation à être diffusée en métropole le CNC doit d'urgence trouver aussi des solutions. Je l'ai dit à l'aune de cette PPL pour assurer une meilleure visibilité en métropole du cinéma ultramarins qui a une très longue histoire pour terminer et pour conclure, je voudrais encore remercié son auteur notre collègue Catherine Conconne car ça PPL touche à une question de justice, à une question d'égalité et de promotion des droits culturels et comme je le disais en introduction, elle est donc une nécessité je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est maintenant à madame la présidente, Éliane. Du groupe pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Pardon monsieur le ministre. Je suis désolé, on m'annonce Monsieur Riester dans les murs. Et donc je souhaiterais si c'est possible une suspension de séance. Quatre minutes.

On ne peut pas attendre tout le Sénat parce que on. Oui enfin bon oui. Écoutez, je ne veux pas vous faire rater votre train et défendra ou d'outre-mer à La Haye. Donc je suspends la séance. Merci monsieur

La séance est reprise. Dans la suite de la discussion générale. Je donne la parole à Madame, la présidente, Éliane Assassi. Pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Cet alors dans l'histoire double annonce pour vous madame la présidente. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a quelques semaines encore, la France a accueilli l'un des plus grands festivals du monde dédié au cinéma, le festival de Cannes. 2 semaines durant lesquelles réalisateur amoureux du cinéma et tant d'autres personnes se rend compte de travail et découvrent de nouvelles Oeuvres pour ainsi donner du sens à ce que représente la culture au quotidien. Et mais Césaire le rappelait bien. La culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort. Ah frontale. On ne peut que souscrire à ces propos que partageait mon regretté ami et camarade Jack Ralite ce poète en politique. Qui ne cessait de rappeler que la culture est un droit. Et un bonheur. C'est donc un devoir de nous assurer de sa transmission. De sons n'accessibilité afin de faire de la culture, un droit essentiel pour toutes et tous. Le Champ de la culture est vaste. Et le cinéma comme d'autres est un art populaire. Or les salles obscures ont été fortement touchés par la crise sanitaire et l'évolution des plateformes numériques les entrées enregistrées avec la avant la crise de de la Covid n'ayant pas repris et cette situation faut autant en Hexagone que et donc c'est dans ce contexte que les distributeurs de films souhaite augmenter le taux de location que les exploitants leur reverse sur les entrées en salle ce taux ça cela a été dit est actuellement de 50% dans l'Hexagone et de 35% dans les outre-mer les distributeurs les plus importants. Je souhaite donc un alignement des taux de location en outre-mer sur ceux de l'Hexagone et les négociations entre les 2 acteurs ont débuté depuis quelques mois. Il est utile, je pense, de rappeler que l'offre culturelle en outre-mer fait face à de nombreuses contraintes. Je le redis aussi puisque ça l'a été dit précédemment par monsieur le le le ministre les coûts d'exploitation et d'investissement sont plus élevés qu'en France métropolitaine pour tenir compte justement des normes sismiques cyclonique et de l'éloignement ou de, ou d'exigences de sécurité propre pour compenser. C'est fort coût, le coût moyen du billet du cinéma est plus élevé. Alors que la fiscalité est moindre. Cette proposition de loi de notre collègue Catherine Conconne que je salue apparaît comme la conclusion d'un échec entre les la négociation dans les négociations entre les exploitants et les distributeurs. La situation est donc préoccupante car elle touche à un principe important et fondamental. La diffusion de la culture. D'un côté les distributeurs justifie cette hausse pour éviter un appauvrissement de l'offre de films, de l'autre les exploitants voit cette dans cette hausse enfin fois cette hausse comme une menace existentielle. Ce sont les populations ultramarines qui vont subir cet échec dans un contexte de crise sociale est aussi rappelons-le à une crise de l'énergie, les prix augmentent partout et les conséquences sont terribles au quotidien. Il est regrettable que la seule issue possible pour espérer que les discussions reprennent soit l'issue législative comme cela été rapport rappelée par Madame la rapporteure. Nous espérons que ce texte permettra d'apaiser le climat et être perçu comme un moyen et non une fin en soi pour que les 2 acteurs qui jouent un rôle essentiel dans l'accès au cinéma puisse trouver une solution qui convienne à tous. Mon groupe et moi-resteront vigilants sur ce sujet sujet des rencontre continueront d'avoir lieu entre mes collègues de la commission de la culture ainsi que les parties prenantes. Notre rôle est d'agir avec responsabilité face à une situation qui risque d'avoir de lourdes conséquences sur la Sid-Ahmed cinématographique en outre-mer et donc c'est le sens de cette proposition de loi qui, espérons-le, sera un levier afin d'apaiser les relations et faire de l'intérêt général. Notre boussole collective pour toutes ces raisons, le groupe CRCE votera en faveur de cette proposition de loi. Merci. Si madame la présidente, avant que je ne donne la parole à Monsieur Pierre-Antoine Levi. Pour le groupe Union. Centriste pour six minutes. Je signale à la Haute Assemblée que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public sur l'ensemble de ce texte et par conséquent, je demande au groupe de s'y préparer. La parole est donc à Monsieur Pierre-Antoine Levi. Pour le groupe Union centriste pour six minutes. Monsieur le président, monsieur le président de la commission culture. Madame la rapporteur, madame l'auteur. Catherine Conconne, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi visant à assurer la pérennité des établissements du spectacle cinématographique et l'accès au cinéma dans les outre-mer. Le cinéma, activités culturelles populaire dans les Outre-mer et structuré autour de différents acteurs principalement privés. Ces établissements ton face à des défis spécifiques, notamment des coûts d'exploitation et d'investissement plus élevés en raison des normes. Sismiques cyclonique de l'éloignement ou d'exigences de sécurité propre. Pour comprendre le contexte il est important de définir ce qu'est un taux de location. Il s'agit du pourcentage du prix de billet qui est reversée par l'exploitant de la salle de cinéma au distributeur du film. En d'autres termes, c'est une part du revenu généré par chaque billet vendu qui revient au distributeur. Historiquement, ce taux est de 35% dans les Outre-mer, où il est appliquée de façon forfaitaire cependant. Liste des distributeurs les plus importants souhaite un alignement des taux de location en outre-mer sur ceux de l'Hexagone qui se situe en moyenne proche du plafond de 50% fixé par le code du cinéma et de l'image animée. Cette augmentation du taux de location serait insoutenable pour les exploitants ultramarins et pourrait aboutir à la fragilisation extrême du secteur ainsi que la fermeture d'établissements laissant certains territoires dépourvus de salles de cinéma. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à plafonner à 35% les taux de location renversé par les exploitants d'établissements cinématographiques ultramarins aux distributeurs de films. Cette mesure permettrait d'assurer la pérennité de leurs établissements et l'accès au cinéma pour les habitants de la dite outre-mer. Il est crucial de noter que cette proposition de loi est soutenue par les exploitants du cinéma d'outre-mer qui ont alerté les parlementaires ultramarins des contraintes économiques pesant sur ces territoires. 12 organisations professionnelles de distributeurs et de producteurs se sont opposés à cette proposition, arguant que restreindre les possibilités de rentabilité de la distribution ne peut pas être la réponse aux difficultés rencontrées par l'exploitation d'outre-mer. Six organisations soutiennent que le plafonnement du taux de location à 35% aurait des effets contre-productifs pour les territoires d'outre- mer eux-mêmes et le public. Cela pourrait peser sur la diversité de l'offre dans les départements et régions outre-mer sur l'accès du public aux Oeuvres et in fine et sur le maintien de l'emploi.

Les coûts d'investissement par fauteuils sont significativement plus élevé qu'en métropole atteignait entre 9500 et 11.000 euros. Comparé à 4500 euros de plus l'éloignement géographique augmente les coûts d'acheminement du matériel. Les normes parasismiques et anticycloniques les charges en électricité due à la climatisation permanente l'usure plus rapide du matériel, du fait de l'humidité et la part importante consacrée à la sécurité sont autant de facteurs qui alourdissent les coûts d'exploitation. Nous pensons qu'il est essentiel de préserver l'accès à la culture dans les Outre-mer et de soutenir les établissements qui font face à des défis spécifiques. Nous devons veiller à ce que les taux de location soit équitable et permettent aux exploitants de continuer à offrir leurs services à la population. Il est également crucial de prendre en compte les conséquences de la crise du Covid-19, qui a forcé les exploitants sur la France entière pendant plusieurs mois, entraînant une perte importante de recettes. Cette situation exacerbé les tensions autour du taux de location mettant en péril la survie des salles de cinéma en outre-mer. Nous devons également considérer le risque que cette situation pose pour le consommateur final. Si le taux de location n'est pas plafonné à 35% les clients pourraient se retrouver à payer la note s'avec des places qui pourrait dépasser les 14 euros. Cela risquerait de réduire encore plus le nombre de spectateurs dans les salles, aggravant la crise du secteur. En conclusion, le groupe de l'Union centriste soutient et votera en faveur de cette proposition de loi convaincu de la nécessité de soutenir le secteur du cinéma dans les outre-mer. Nous pensons qu'il est essentiel de maintenir un taux de location équitable qui tienne compte des défis spécifiques auxquels sont confrontés les exploitants du cinéma en outre-mer. Nous devons veiller à ce que le cinéma reste accessible à tous indépendamment de leur lieu de résidence. Je vous remercie.

Monsieur le. Monsieur le ministre, madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. La lettre de, de constitution prévoit que la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture ce principe plus que jamais nécessaire à notre temps est énoncée à l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946. Tout le monde ne peut pas aller facilement à l'opéra ou au Louvre. Il est des arts dont beaucoup non que la reproduction un enregistrement une photographie une retransmission. Il en est d'autres dont on peut plus aisément faire une expérience in altéré. Voir un film à Cannes ou à Cayenne, c'est la même expérience. L'oeuvre est la même et cette expression culturelle authentique est accessible. Cette accessibilité mérite d'être soutenu la diffusion de la culture doit être assurée autant en France métropolitaine. Quand outre-mer. La proposition de loi que nous examinons fixe le plafond du taux de location à 35% dans certains territoires d'outre- mer contre 50% actuellement. La situation des établissements de cinéma ultramarins diffère de celle des établissements de métropole à plusieurs égards. Tout d'abord ceci repose sur un équilibre économique particulier caractérisé par des marchés plus restreints et des coûts d'exploitation et d'investissement plus élevé, dû notamment à la mise en conformité face aux risques naturels. Pour ces raisons, la rentabilité de ses de ces établissements est plus faible qu'en métropole malgré une taxation avantageuse et un prix du billet plus élevé. Une autre différence notable concerne le taux de location qui est l'objet de la présente, proposition de loi. du prix du lait, du prix du billet qui est reversée au distributeur du film que celui-ci négocie avec l'exploitant d'établissement du de cinéma. Actuellement, le droit fixe cette part entre 25 et 50% de la base film. Historiquement, le taux de location et de 35% d'outre-mer compte 47% environ en métropole cette différence entraîne néanmoins un écart de recettes relativement faible pour le distributeur. En effet, du fait de la fiscalité réduite applicable en outre-mer associé à un ticket plus coûte en moyenne pour une place de cinéma. Le distributeur perçoit 2 euros 70 en outre-mer. Contre 2 euros 78 en métropole. Lors de récentes négociations cependant les distributeurs ont émis le souhait d'aligner le taux de location ultramarins sur celui de la métropole. Tout en reprenant la charge de la distribution locale jusque-là assurée par un intermédiaire spécialisé. Les exploitants ultramarins redoutent qu'une telle hausse force. Nombre d'entre eux à mettre la clé sous la porte du fait de leur contrainte financière particulières et des conséquences encore perspective de la crise sanitaire sur la fréquentation des cinémas. De leur côté les distributeurs avancent également les difficultés liées à la pandémie et estime que la fixation d'un plafond à 35% grèverait leurs chances de rentabilité. Il deviendrait dès lors plus frileux, ce qui pourrait attention in fine et entraîné un approuveraient Isman de l'offre en outre-mer et donc une baisse de l'accessibilité des Oeuvres cinématographiques. On peut donc on peut malgré tout douter de cet argument parce que cette situation serait davantage le résultat d'un rapport de force déséquilibré qu'une conséquence inévitable. Les Les enjeux financiers est en réalité limitée pour beaucoup de distributeurs. Je crois que l'expression l'exception culturelle française prend aujourd'hui tout son sens dans la défense d'un égal accès à la culture sur l'ensemble de notre territoire. L'égalité, c'est pas l'uniformité et les politiques publiques doivent prendre en compte les différences. Au sein de notre commission, nous partageons l'espoir que cette discussion donnera un nouveau souffle aux négociations entre les différents acteurs. C'est pourquoi le groupe RDSE. Votera cette proposition de loi.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Cette proposition de loi traite d'une question spécifique au territoire outre-mer de l'article 73 de la Constitution soit la Guadeloupe la Réunion la Martinique la Guyane. Et Mayotte. Elvis 21 établissements actifs en 2022 dans certains comporte plusieurs salles. Sur ce territoire plus encore qu'ailleurs, les salles de cinéma sont un vecteur essentiel de divertissement populaires d'ouverture au monde et de socialisation. La crise sanitaire a pu faire craindre avec l'effondrement des entrées une mise en danger de l'exploitation des films en outre-mer d'autant qu'une partie du public a découvert les usages des plateformes durant la crise. En outre-mer, mer comme en métropole. Le public a cependant regagner les salles confirmant et nous nous en réjouissons la solidité du secteur. Je citerai les récents travaux de la mission d'information sur la situation de la filière cinématographique en France dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteure avec mes collègues Sonia de la Provôté, Jérémy Bacchi. Notre rapport intitulé Le Cinéma contre-attaque entre résilience et exception culturelle un art majeur qui a de l'avenir, analyse le succès du cinéma français, de la fréquentation de nos salles. Nous avons identifié trois atouts majeurs. Tout d'abord la richesse et la diversité de l'offre de films. Deuxièmement, un succès populaire jamais démenti, et enfin une structuration de la filière dans laquelle les financements publics compte pour un quart et c'est une véritable exception culturelle française. Dans ce paysage, la diffusion des films en outre-mer comporte plusieurs particularités, le niveau des charges d'exploitation est plus élevé. Notamment le respect des normes anti-cyclonique et para-sismique, l'usure des matériaux provoquée par un climat humide, les contraintes liées à l'éloignement des salles entraîne des coûts spécifiques. La sécurité est également un poste important pour les exploitants de salles. Elle représente en moyenne 10% du chiffre d'affaires des salles ultramarines, contre environ 1% en métropole. En raison de ses contraintes financières, les territoires Outre-Mer bénéficient d'avantages fiscaux. Une TVA plus faible qu'en métropole, ainsi qu'une taxe allégé sur les prix des entrées aux séances la TSA. D'autre part et cela fait l'objet de cette proposition de loi, les salles bénéficient d'un taux de location plus avantageux qu'en métropole. Cela a été dit, le taux de location des films dits au distributeur par l'exploitant de la salle représente historiquement 25% du chiffre d'affaires de ce dernier. Ce pourcentage fluctue au contraire en métropole où il est aujourd'hui de 47% en moyenne. Cette différence, fruit d'un consensus d'une cinquantaine d'années est remise en cause par les distributeurs. Il souhaite un alignement du taux sur celui pratiqué en métropole, faisant valoir leurs difficultés financières suite à la crise sanitaire et une différence de traitement qui leur paraît aujourd'hui injustifiée. Ils invoquent également les coûts engendrés par le récent passage à une distribution directe. Notre rapporteur Sylvie Robert dont je tiens à souligner la qualité du travail. Rejetant tout a priori relativise cependant la portée de cette différence de traitement. La position des distributeurs semblant tête surtout une question de principe. Les exploitants de films quant à eux estiment qu'elle ne pourrait pas faire face à une augmentation du taux de location qui remettrait en cause leur viabilité. Il faut souligner que, malgré les elle le prix du billet en outre mer reste sensiblement plus élevé qu'en métropole, augmenter le taux de location conduirait à augmenter encore le prix du billet, ce qui risque de devenir dissuasif pour les familles dans un contexte déjà inflationniste. Les auteurs de la présente, proposition de loi sont intervenus pour éviter les conséquences de l'alignement des taux sur la diffusion et la diversité des films en outre-mer je pense que les intérêts ultramarins impose en effet pour le moment un plafonnement du taux de location à 35%. Afin d'éviter la mise en danger de l'équilibre économique du secteur. Il s'agit d'ailleurs de la recommandation figurant dans un rapport de l'inspection des finances de 2018. Je tiens à souligner également que notre intervention législative se justifie par l'absence de conciliation des acteurs. En présence, car je le rappelle, des négociations menées à l'initiative du CNC n'ont pas abouti. À l'image du rapporteur. Nous souhaitons une reprise de ces négociations commerciales dans un climat apaisé qui est dans l'intérêt de tous et surtout du public ultramarins dans cette attendent notre groupe apportera son soutien au texte. Je vous remercie. La parole est maintenant Monsieur Jean-Pierre Grand. Pour le groupe les indépendants pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La crise sanitaire a fait mal aux exploitants des salles de cinéma partout en France, la fréquentation a beaucoup baissé et n'a globalement toujours pas retrouvé son niveau d'avant la crise, même si la fréquentation sur le mois d'avril 23 a été excellente, les outre-mer comme l'Hexagone font face à ces difficultés. Mais pour les territoires ultramarins d'autres problématiques s'ajoute, je ne reviendrai pas sur l'explication du mécanisme de par la répartition du prix d'un billet de cinéma dans ces territoires, cela a été très techniquement et surtout reviens fait. Par la rapporteure du texte. Il ressort ainsi de ce mécanisme. Que la base film du billet est une plus élevé dans les Outre-mer qu'un hexagone pourtant l'équilibre économique des établissements de cinéma ultramarins et plus largement l'accès à cette activité. Culturelle sont menacés. Il en est de même pour le prix des billets de cinéma qui est en moyenne plus élevée dans les Outre-mer. Cela pose déjà en soi une la question de l'accès à cette activité populaire et familiale dans des régions dans lesquelles le pouvoir d'achat de nos concitoyens et déjà mis à mal par des prix plus élevés que dans tous les secteurs de la vie quotidienne, Les exploitants de salles s'il bénéficie certes d'avantages fiscaux doivent en revanche composer avec les marges très très étroite et des coûts d'exploitation investissements plus importants afin de respecter les normes sismiques ou cyclonique. Malgré une base de films plus importants. La rentabilité économique des établissements restent donc difficile à atteindre et à certains et certains sont déjà en danger. À cette situation précaire s'ajoute aujourd'hui une nouvelle contrainte, la menace de l'augmentation du prix de location renversé par les exploitants d'établissements aux distributeurs de films, ce taux est actuellement plafonné à 50% pour toute la France, sans distinction entre l'Hexagone et outre-mer mais il se situe en pratique, autour de 35% dans les territoires ultramarins une augmentation du prix pourrait conduire à la fermeture de certains établissements. Dans ces régions qui ne quand déjà pour la plupart que peu d'établissements n'en compte que trois en Martinique, seuls à Mayotte par exemple assurer leur pérennité est essentiel, c'est justement l'objet de cette proposition de loi qui vise à plafonner à 35% le taux de location dans les départements et régions d'outre- mer on peut regretter que les négociations distributeurs, exploitants soient révélées infructueuses et que nous devions légiférer sur ce sujet mais comme l'a souligné la rapporteure en commission cette PPL n'est qu'un exemple supplémentaire de la nécessité d'adapter le droit aux spécificités ultramarines. Qui sont nombreuses. qu'il serait aussi bien souvent pertinent de tenir compte des spécificités entre les outre-mers. Les outre-mer nous partageons l'objectif de cette proposition de loi qui vise à aider les exploitants de salles et à garantir l'accès des ultramarins au cinéma. Nous espérons toutefois vivement qu'elle ne mènera pas un appauvrissement de l'offre cinématographique dans dans les Drôme. En conduisant certains distributeurs à déserter leurs salles de cinéma au motif que le plafonnement du taux de location ne leur permettait pas de couvrir leurs frais, cela serait préjudiciable aux ultramarins à l'opposé de l'objectif de cette proposition. Nous espérons donc l'adoption de ce texte que nous souhaitons relancera les négociations entre les distributeurs les exploitants de façon raisonnable et raisonnée et notre groupe naturellement votera ce texte. Merci, cher collègue, la parole est maintenant madame Monique de Marco pour le groupe écologiste pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure madame l'auteur. Mais c'est mes chers collègues. Parlons tout d'abord des salles de cinéma. Ce ne sont pas seulement des salles obscures. Ce sont aussi des salles de fraîcheur ou les passants vont se réfugier pendant les vagues de chaleur. Des propositions émergent d'ailleurs pour pratiquer des tarifs réduits en période de canicule, comme l'a proposé dans son rapport, le Conseil de Paris, Paris à 50 degrés. Dans les territoires ultramarins. Pays de la saison unique selon Édouard Glissant romancier philosophe martiniquais. La climatisation des salles il est permanente. Cette différence climatique explique l'énorme différence de coûts d'investissement par fauteuil. Il faut rajouter le respect des normes para-sismiques anticyclonique ou encore l'usure du matériel lié au taux d'humidité. Des plus élevés. Les coûts d'investissement, ils sont de ce fait plouk 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone jusqu'à 11.000 euros compte 4500 euros dans l'Hexagone. C'est pourquoi depuis 50 ans les exploitants, les exploitants de salles ultramarins bénéficie d'un taux de location, plus faible que dans la France hexagonale. 35% de taux de location quand 46% en moyenne. Cela est aujourd'hui remis en cause par les distributeurs de films, essentiellement basés hors de ses territoires qui demandent un alignement sur les Cela intervient aussi après le contournement des intermédiaires locaux par des distributeurs hexagonaux. Pour une distribution dite en Direct. Dans le même temps la forte inflation à réactiver la question du coût de la vie dans les territoires ultramarins. Une commission d'enquête a été créée à l'Assemblée nationale pour enjoindre le gouvernement de réagir alors que la dernière étude sur le différentiel des prix consacré à l'Outre-mer de l'Insee date de 2015. On pourrait appliquer l'analyse générale de son rapporteur au secteur du cinéma. Les exploitants de salles, ils subissent aussi une forme de captivité économique. À contrario, les distributeurs, avec qui il traite établissent leurs mars sur l'ensemble du territoire national. Les exploitants sont attachés à leur territoire, ils ne peuvent pas ajuster leur activité oxyde de ces aléas. Ce fut particulièrement le cas pendant le Covid. Les territoires ultramarins ont également été plus durement touchés par la crise sanitaire. Ce qui s'est répercuté sur la fréquentation des salles. Selon le bilan d'activité du CNC pour 2022 la fréquentation, ils seraient toujours en recul de 32,1% par rapport à la moyenne 2017 2019. qu'on leur forte concentration en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique Iran leur survie essentiel. Nous soutenons donc cette proposition de loi de Catherine Conconne qui offre une solution pour garantir le prix des places, dont l'accès au cinéma dans les territoires visés par l'article 73 de la Constitution. À long terme. Le goût de la salle continuera de faire naître je l'espère de nouvelles vocations dans les territoires disposant de tous les atouts pour attirer les tournages. La formation des jeunes soit 6 renforcée en appui avec les régions et le CNC. Cela s'inscrit également dans la logique de l'aide sélective du CNC intéressant les cultures d'Outre-mer. À quoi bon, soutenir le développement du film. Si les salles mettent la clé sous la porte. Nous ne pouvons qu'encourager l'accès à la culture cinématographique qui passe par le maintien d'un tarif raisonnable. En espérant que les négociations hein très exploitant distributeur puis être puissent être relancé prochainement dans l'intérêt de toutes et tous, nous voterons bien évidemment pour cette proposition de loi. Merci cher collègue. La parole est maintenant monsieur Thani Mohamed Soihili pour le groupe RDPI pour 4 minutes. minutes. Le président, Monsieur le Ministre ce président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Le cinéma est un art qui transcende les frontières, les langues et les cultures. Il permet de nous divertir de nous émouvoir de réfléchir et de nous connecter aux histoires du monde entier. Il est essentiel que tous les citoyens qu'il réside dans un Hexagone ou dans les territoires d'outre-mer et accès à une programmation cinématographique variée et de qualité. Cependant, un outre-mer cet accès est souvent limité, voire inexistant. À Mayotte, par exemple, il n'existe que deux Établissements qui hein diffuse dont le fonctionnement n'est pas régulier de surcroît. Entre géographie norme spécifique lié au phénomène climatologique ou géologiques, prix du billet plus élevé pour tenir compte de charges de contraintes d'exploitation spécifiques les cinéma d'outre-mer sont particulièrement fragilisés. Cela crée un fossé culturel inacceptable et limite les opportunités de développement artistique et économique local. En plus de ces difficultés, les distributeurs de films pèsent de tout leur poids pour aligner le taux de location de leurs films sur celui pratiqué dans l'Hexagone afin de le faire passer de 35 à 50%, c'est David contre Goliath et la mort assurée de nos établissements. Si nous ne faisons rien car, de fait, une telle mesure aurait inévitablement des répercussions sur la rentabilité de ces salles de cinéma qui verraient leur fragilité économique s'accroître dans une période déjà marquée par les conséquences de la crise du Covid et une inflation importante. Et se traduirait un autre par une hausse du prix du ticket qui accentuerait le risque de désintérêt des salles de cinéma au profit des plateformes numériques et mécaniquement par une fermeture définitive de ces établissements. Pourtant le cinéma qui combat l'oisiveté est un facteur de cohésion sociale, je pense à mon département et aux enjeux particuliers auxquels il est confronté. La fermeture d'un lien de divertissement, alors qu'il n'en existe pas suffisamment sur place serait délétère. Aussi le groupe RDPI soutiendra vivement la présente, proposition de loi qui vise à plafonner à 35% les taux de location reversés par les exploitants d'établissements cinématographiques ultramarins au distributeurs de films. Je remercie à ce titre, notre collègue Catherine Conconne d'avoir pris l'initiative de cette proposition de loi et je sais gré au gouvernement d'avoir su comprendre l'urgence de la situation en engageant la procédure accélérée. Je profite de mon intervention pour pousser plus en avant la réflexion autour du cinéma ultramarins. Tout à l'heure, le ministre des Outre-Outre-mer nous préciser des mesures prévues pour soutenir financièrement les établissements de spectacles cinéma photographique dans nos régions d'Outre-mer. Des investissements. Essentiels sont de nature à maintenir la qualité des salles de cinéma, et à améliorer l'expérience globale pour les spectateurs. Il faudrait également accentué des dispositifs de soutien à la création et à la production cinématographique locale. Il m'apparaît primordial de favoriser l'émergence de talents locaux de renforcer la visibilité de cinéastes ultramarins et de favoriser le rayonnement sur la scène nationale voire internationale et de promouvoir la diversité culturelle à travers des films reflétant la réalité et les spécificités de ces territoires en définitive ah soutenant unanimement cette proposition de loi. Nous envoyons un message clair, l'accès au cinéma est un droit fondamental, qui ne devrait pas être limitée par notre géographie. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire une réelle différence dans la vie des habitants des Outre-mer et de prévenir, notre Patrimoine culturel. de préserver notre Patrimoine culturel. l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi, je vois. Appel que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Votants 342. Exprimés. 341. Pour 341. Contre 0 la proposition de loi est adopté à l'unanimité. Je félicite Madame Conconne. C'est assez rare dans cet hémicycle. Donc bravo. Merci à vous. Oui madame Cohen. Vous voulez dire quelques mots bien entendu. Merci monsieur le président, Monsieur le mini, chers collègues. Je tiens à remercier cette belle unanimité qui a présidé au vote de la proposition de loi qui tend à garantir l'existence de nos cinémas je tiens vraiment du fond du coeur à vous dire merci savez le grand poète a dit. Tous les hommes ont des devoirs mais du lot commun il y en a qui ont plus de voix que d'autres. C'est ce sens du devoir qui me fait tous les jours me battre au quotidien tous les jours dans cet hémicycle pour réclamer en permanence plus d'équité et un prisme de regarde totalement différent sur nos pays. À cette république qui entend qui comprend et qui s'accommode désormais de sa bienfaisante diversité cette république qui fait honneur et qui devra faire honneur plus que jamais à la notion d'équité, de solidarité et de ce sens légitime de la nuance cette république qui doit protéger aussi enfin j'ce mot pour le dire. Les distributeurs le lien ne doit pas se couper fait au mieux pour vous accommoder de nous de nos évidences et de nos réalités, cette loi n'est pas une loi contre vous un seul principe désormais devrait présider à ses relations c'est celle des vertus républicaines que j'ai évoquées notre dénominateur commun, la culture. Devrait, comme l'a souhaité aussi le poète rendent nos vies vivable. C'est tout le bonheur que je souhaite à tous. Merci madame qu'on connaît et tout le monde reconnaît votre passion dans cet hémicycle. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport, présenté par monsieur Sébastien Pla et plusieurs de ses collègues, à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Sébastien Pla, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes.

Monsieur le. Le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission culture éducation monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Nous avons la liberté de croire qu'en ce jour du 15 juin 2023. Nous pouvons par notre voix donner un signe fort en amplifiant la lutte contre le fléau des agressions sexuelles sur mineurs aujourd'hui. Nous avons la volonté d'affirmer que nous, nous voulons plus un seul pleure plus haut que sanglots plus aucune larme de honte sur les joues d'un enfant qui est pratique une activité sportive. Nous voulons des larmes de joie des étoiles dans les yeux des émotions que seul le sport Cécilia nous procurer. Les enfants, mes chers collègues, nos enfants. Nous avons le devoir de les protéger de leur permettre de s'épanouir sans entrave aucune à l'accomplissement de leur humanité. Tous les enfants méritent que nous leur prêtions attention et il est parmi eux trop d'enfants qui souffrent et que l'eau n'entame pas. Qui ne parlent pas et qui peut être ne parleront jamais de leur enfance volée. Portant un silence lourd fardeau qui après avoir détruit leur corps à briser leur rame. Écoutons les témoignages rendus publics ce des victimes de la pédophilie, écoutons leurs exigences de justice. 75% des enfants connaissent leurs agresseurs mais peu osent les dénoncer par peur de représailles, et surtout par honte. La pratique sportive fournit un terreau favorable à l'apparition de ces violences. Les contacts physiques souvent nécessaire le dépassement de soi sont autant de situations à risques. Tout comme l'écosystème de la pratique sportive, les vestiaires, les douches le covoiturage. Les stages à internat ou encore les son effectif festives sont autant de lieux où les prédateurs chassent leurs proies vulnérables prise au piège. Le Leadership autoritaire peut déséquilibrer le rapport de force entre les entraîneurs et les athlètes et ce d'autant que le sport. Le jardin masculin prédomine et peut conduire à des abus de position dominante et que c'est un milieu où les incidents sont facilement étouffée et où l'omerta prédomine cette difficulté à assumer son état de victimes. Et à le faire reconnaître. Sarah Abitbol 10 fois championne de France et médaillé de bronze aux Jeux olympiques et mondiaux femme courageuse. La portée du durant 30 longues années. Il a fallu du temps pour que ce silence, silence se brise que l'omerta soit rompu. Oui il y a eu un avant et un après Sarah Abitbol, un de ces témoignages qui font boule de neige, puisque le témoignage de Sarah a entraîné 200 athlètes dans son sillage dans près de 40 fédérations de différentes. Non, ce n'était pas elle la coupable, le coupable c'était son entraîneur cette personne de confiance. Celui dont je cite les propos de Sarah ont redouté par ses colères son charisme, sa violence durant les entraînements à nous projeter au sol celui. Qui, mes parents avaient toute confiance pour m'accompagner après les entraînements, lui qui prétendait me faire travailler davantage quand j'avais mauvais caractère. Lui qui demandait à Sarah de terre ce lourd secret. Un mécanisme d'emprise bien rodée régulièrement décrit par les sportifs qui ont accepté de se confier. Et pourtant malgré ces témoignages. Seuls 40% des victimes pour mener leurs agresseurs jusqu'au procès, suivi d'une condamnation. Pourquoi. Par le fait de la prescription bien sûr mais aussi parce que les victimes. Honte honte ont peur de porter une vie durant le fardeau de ce silence, grâce au courage de ces athlètes et aux témoignages poignants de Sarah Abitbol. Le mouvement de libération de la parole à gagner le du sport pour que la honte et la peur puisse changer de camp. Mes chers collègues. Ce texte, que nous allons examiner, c'est la proposition de loi Abitbol. Que je porte avec beaucoup d'émotion d'humilité, de pudeur et avec un profond profond engagement je sais pouvoir compter sur vous tous et vous toutes mes chers collègues je sais pouvoir compter sur vous, madame la Ministre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en appelle à cette chambre pour que nous puissions travailler de concert pour sanctuariser plus encore le milieu du sport afin que les enfants soient en sécurité afin que chaque parent puisse se confier son enfant sans crainte et que cela permette surtout de lever tout soupçon qui pourrait planer sur les clubs dans ma quête de la compréhension du phénomène. J'ai été très souvent bouleversés par le récit glaçant des victimes. J'ai été le témoin indirect des souffrances qu'elles ont enduré ces témoignages d'une violence inouïe, d'une telle perversité. Touché au plus profond de mon âme. J'ai rencontré des dirigeants de clubs qui parfois n'ont pas pris la mesure du fléau cherchant à minimiser, souvent par méconnaissance des mécanismes utilisés par les prédateurs. Mais nombre d'entre eux ont conscience que tout cela est inacceptable et s'engage à lutter contre les violences sexuelles mais reconnaissent se trouver démunies par manque d'information, de formation et surtout de temps. Pas pointant les contraintes et les limites du bénévolat. Dans les faits, on estime que près d'un sportif sur sept déclare avoir fait l'objet d'atteinte à son intégrité. Il n'y a pas une semaine sans qu'un témoignage d'agressions sexuelles ne soient rendues publiques. Nous devons agir en amont pour couper l'herbe sous le pied des prédateurs. La lutte contre les violences sexuelles est un aveu. que nous devrons gravir, pas à pas, c'est aux propositions de loi n'est comme pas de plus permettant d'améliorer les dispositions existantes de protection des mineurs en renforçant l'incapacité d'exercer des potentiels prédateurs accompagnant Madame la Ministre dans son combat pour le sport éthique et en particulier contre les violences sexuelles. Déjà en 2019, l'émission la mission d'information sénatoriale sur la prévention, la détection et la répression des infractions sexuelles sur les mineurs conduite par nos collègues Catherine Deroche et Michelle Meunier appelé à un renforcement du contrôle de l'honorabilité des adultes en contact avec les enfants en. Partout les standards les plus hauts. La loi de 2021, confortant le respect des principes de la République a complété le Champ des personnes soumises au contrôle d'honorabilité dans le sport au côté des encadrants éducateurs sportifs professionnels les éducateurs sportifs bénévoles sont désormais soumis à l'obligation d'honorabilité. Ah c'est faire le système d'information automatisés des personnes concernées. Disposant d'une licence a été mise en place. Pourtant, force est de constater qu'il demeure des situations où des adultes sont placés en contact des enfants sans qu'il ne soit réellement contrôlés sans qu'ils aient fait preuve de leur honorabilité. Je propose d'inverser la charge de la preuve qui pèsent actuellement sur les victimes. Ah la faisant porter sur les adultes. Qui doivent attester de leur honorabilité dès lors qu'ils sont en contact avec des mineurs. Je souhaite que l'on puisse s'assurer que ce contrôle hé bien opéré mais aussi responsabiliser l'ensemble des acteurs du monde sportif en incitant chaque club à prendre une part active dans la prévention et ainsi éviter d'exposer les enfants à des risques qu'on pourrait mieux anticiper. Que les agresseurs se sentent visés. Traqué, qu'ils sachent que les adultes forment autour des enfants une chaîne solide de contrôle et de protection. Je veux saluer le travail de notre collègue rapporteur Jean-Jacques Lozach, qui a su ménager les ambitions d'un texte visant à renforcer les contrôles qui pèse sur les adultes et le nécessaire besoin de préserver le bénévolat dans les clubs et associations. Ce texte ressort enrichi des auditions conduites du débat parlementaire en commission et en collaboration étroite avec les services du ministère, c'est une avancée collective. Transpartisane que je tenais à saluer au service d'une cause universelle, un texte construit dans l'échange et avec la volonté d'agir d'agir vite. Les membres de la commission compléter ce dispositif proposé en renforçant le régime d'incapacité et l'obligation pour les dirigeants de clubs de signaler les comportements à risque, sauf à s'exposer eux-mêmes à des sanctions pour lesquels les préfets disposeront de moyens coercitifs nous propose aussi d'introduire dans le Champ sportif. Le renforcement du contrôle d'honorabilité dont a bénéficié le secteur social et médico-social par la loi, attaquée en 2022. À savoir le fait qu'une inscription d'une condamnation jaillissent maintiennent à l'incapacité d'exercer. Même si la condamnation a disparu du casier judiciaire B2 de la personne ne doute. Preuve année que la cible touchée et juste. Les auditions ont révélé que la par la cellule ministérielle qui recense depuis 2021 les violences sexuelles dans le sport que sur la moitié des éducateurs et licenciés bénévoles contrôlé soit un million. D'éducateurs encadrent licencié bénévoles 440 incapacité ont déjà été notifiées épreuve années qu'il est nécessaire d'ajuster les choses pour arriver à contrôler chaque année l'intégralité des 2 millions d'éducateur bénévole licenciés. Je prends contact des améliorations proposées à l'unanimité par la la commission culture et éducation et miennes au cours des auditions de sportifs et associations de victimes Tous ont insisté sur la nécessité d'impliquer plus encore les clubs. Je suis intimement persuadé que c'est au quotidien dans les clubs en sensibilisant les acteurs du terrain placés au contact des jeunes sportifs que l'on trouve l'une des clés de la réussite de notre combat. C'est pourquoi, au-delà de ce texte au-delà de l'engagement républicain entre l'État et les fédérations. Il nous faut étudier l'opportunité de créer un référent intégrité par club. Il serait en contact étroit avec la cellule signa sport formés pour mieux détecter prévenir les gestes et pratiques à risque est chargée de recueillir la parole des victimes, puis le cas échéant signaler tout comportement déviant auprès des instances compétentes et de l'administration. Je voudrais remercier vivement l'ensemble des sportifs, artistes, représentants d'associations de victimes qui, par leur initiative ont publié une tribune ce matin à l'équipe de soutien soutiendront et qui nous apporteront tout le soutien pour continuer à lutter contre les violences sexuelles dans le milieu sportif. Enfin, je vous propose madame la Ministre. A cette année de Coupe du monde. De rugby à l'approche des Jeux olympiques. De décréter la lutte contre les violences sexuelles dans le sport comme une grande cause internationale en demandant aux équipes de France de porter sur leur maillot la marque de cet appel. Mes chers collègues. Soyons dignes devant la souffrance de toutes ces sportive et de toutes ces sportifs victimes soyons dignes devant le courage à briser le silence, montrant l'engagement fort de la France au reste du monde et élu Tom pour que la honte change définitivement de Camp Mercier. Merci cher collègue. La parole est maintenant Monsieur Jean-Jacques Lozach, rapporteur de la commission de la culture de l'éducation, de la communication pour 10 minutes, 10 minutes et pas 10 minutes 30.

dressait un terrible constat je cite le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles est un dispositif aléatoires et insuffisants qui présente des failles exploitables par les auteurs des violences sexuelles, 90% des éducateurs sportifs ne faisait l'objet que d'un contrôle très partiel dans un secteur où l'omerta a régné pendant longtemps. Néanmoins, on constate un tournant depuis quelques années du fait d'une triple action. De la part du mouvement sportif, tout d'abord, où les révélations de plusieurs athlètes de haut niveau comme Sarah Abitbol ont fait l'effet d'un électrochoc. De la part du ministère. Ensuite, je pense au volontarisme de l'ancienne ministre Roxana Maracineanu nous sur ce sujet volontarisme confirmé depuis. En 2020, le ministère a mis en place une cellule de signalement de faits de violence depuis son lancement, ce soit ainsi, puis de 9107 signalements qui ont été réalisés conduisant à 424, interdiction d'exercer. Vous-même Madame la Ministre venait de lancer un comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport co- présidée par Marie-George Buffet, Stéphane Diagana dans l'une des missions et la protection renforcée des pratiques 40 et des pratiquants, notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination. Le législateur et plus particulièrement le Sénat a posé les jalons législatifs, d'un contrôle renforcé. Nous avons un s'est introduit dans la loi confortant les principes de la République, la loi d'août 2021 l'obligation pour les clubs sportifs de relever l'identité complète des personnes susceptibles d'être éducateur sportif ou d'intervenir auprès des mineurs. C'est un préalable indispensable à la mise en place d'un contrôle automatisé de l'honorabilité des éducateurs sportifs en quelques mois les progrès réalisés sont notables. La mise en place de ce système en lien avec les clubs et les fédérations qui en sont des rouages essentiels a déjà permis de vérifier l'honorabilité de la moitié des éducateurs sportifs. Certes le système reste perfectible et demande en ces premiers mois un travail considérable aux fédérations. Mais regardons le chemin parcouru. Nous sommes passés de contrôles aléatoires et restreint en 2021 à 500.000 éducateurs sportifs contrôlés fin 2022 et à 1 million en mai 2023. Une fois les problèmes informatiques réglé et les bonnes pratiques dans la transmission des noms intégré ce contrôle sera bientôt routinier. La proposition de loi de notre collègue Sébastien Pla renforce la protection des mineurs et le contrôle de l'honorabilité dans le sport. Je salue cette initiative qui permet de combler certains trous dans la raquette. Elle prévoit notamment la vérification de la capacité des éducateurs sportifs à la fois au regard du Fijais, c'est-à-dire le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du bulletin numéro 2 du casier judiciaire qu'on appelle le B Je tiens à souligner des échanges très constructifs que j'ai pu avoir avec le mouvement sportif, ainsi qu'avec vos services madame la Ministre, dans le cadre de la préparation de ce texte. Nous partageons tous au même objectif, lutter contre les violences notamment sexuelles dans le milieu sportif à mon initiative, la commission de la culture a réécrit le texte avec un triple objectif. Alléger responsabilisés. Nous avons tout d'abord aligné les modalités de contrôle des éducateurs sportifs sur celle applicable dans le domaine social et médico-social pour les personnes qui encadrent des publics fragiles. Celles-ci ont en effet été renforcés par la loi relative à la protection des enfants de février 2022, dite loi. Le texte prévoit notamment par exception au principe de réhabilitation pénale. Le fait que l'inscription d'une condamnation au Fijais entraîne une interdiction d'exercer. Même si cette condamnation n'est plus inscrite sur le B de certaines condamnations peuvent en être effacée des 6 mois après le prononcé de la peine à la demande de la personne condamnée elle reste cependant inscrite au Fijais au minimum 20 ans. Les faits commis lorsque la personne était mineur est également inscrit pendant 10 ans. Ce nouveau dispositif répond à une attente forte des fédérations et des services déconcentrés du ministère. Ils sont actuellement confrontés à des contentieux lorsqu'il souhaite, écarter un éducateur sportif inscrit au Fijais mais dont le bulletin numéro 2 du casier judiciaire ne mentionne plus la condamnation comme l'exception au principe de réhabilitation pénale n'est actuellement pas prévu pour le domaine sportif. Certains de ces éducateurs contestent leur incapacité d'exercer selon les informations qui m'ont été transmises plusieurs arrêtés d'interdiction d'exercer pour des personnes inscrites au Fijais ont été annulées par la justice nous complétons également les listes des incapacités en interdisant d'exercer la fonction d'éducateur sportif aux personnes condamnées à l'étranger pour des faits qui commis en France aurait entraîné cette même incapacité. Nous inscrivons aussi dans la loi le principe d'un contrôle annuel de l'honorabilité. Deuxièmement nous avons alléger les obligations pesant sur les dirigeants des clubs. Le texte initial le faisait porter la responsabilité du contrôle du bulletin numéro 3 du casier judiciaire du futur éducateur sportif. Nous avons supprimé cette obligation pour plusieurs raisons. Le contrôle de l'honorabilité doit rester une et prérogatives régaliennes. Par ailleurs, tant les fédérations que le ministère nous ont alerté sur un risque d'alourdissement des charges pesant sur les présidents de clubs dans un contexte de crise du bénévolat. d'ailleurs, d'ailleurs à saluer l'engagement des millions, des milliers de bénévoles qui rendent possible la pratique sportive sur l'ensemble du territoire. En fin de bulletin numéro 3 n'est pas exhaustif, il ne comprend que les condamnations les plus graves, un dirigeant du club pourrait de bonne foi à la consultation de l'extrait judiciaire transmis par l'éducateur sportif penser que celui-ci remplit les conditions d'honorabilité sans que cela soit juridiquement le cas. Nous souhaitons cependant responsabiliser les dirigeants en instaurant l'obligation de signaler au préfet des comportements au sein de leur club présentant un danger pour les sportifs, je pense notamment aux agissements déviants, d'un éducateur. Si les présidents de clubs ont le réflexe de prévenir le procureur. Certains sont réticents à en faire de même avec l'administration, en l'absence de base légale. Or le préfet dispose de pouvoirs de police lui permettant d'écarter rapidement une personne potentiellement dangereuses. Par ailleurs, nous luttons contre des dirigeants qui pourrait fermer les yeux sur les violences commises dans leur club, ils pourront désormais être sanctionné. Nous créons une nouvelle sanction administrative d'interdiction de diriger un club sportif. Il existe aujourd'hui un vide juridique. Alors que le préfet il peut prendre une mesure administrative d'interdiction d'exercer pour les éducateurs sportifs potentiellement dangereux. Il n'existe aucune interdiction similaire pour les dirigeants du club. Le préfet dispose seulement de la faculté de fermer administrativement l'établissement sportif. La sanction administrative que nous créons pourraient être prises dans 3 cas. Lorsque le comportement même du dirigeant de club fait porter un risque pour les sportifs lorsqu'il emploie au maintien en emploi un éducateur sportif, frappé de l'incapacité d'exercer ou enfin lorsqu'il refuse d'informer le préfet de comportements déviants, au sein de son club. Les premiers jalons d'une meilleure prévention des violences contre les sportifs et d'une protection renforcée des mineurs ont ainsi été mises en place. Cette proposition de loi permet de les compléter. Elle est à, elle est attendue par tout le mouvement sportif. Je vous remercie. La parole est maintenant à madame Amélie Oudéa-Castéra Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Vous avez la parole madame la Ministre. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires culturelles de l'éducation et de la communication. Cher Laurent Lafon, monsieur le rapporteur. Chers Jean-Jacques Lozach Monsieur le sénateur cher Sébastien Pla mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Un enfant sur 7 en effet victime de violence dans le sport et derrière ce chiffre effrayant. Combien d'enfants en souffrance dont l'existence a été abîmé, et la vie parfois brisée. Voilà pourquoi notre 1er devoir en tant que responsable publics et de regarder ces violences avec lucidité. Oui, elles prennent des formes diverses, qu'il faut dénoncer clairement pour en faire prendre conscience, violences physiques, psychologiques, harcèlement agression en emprise ou encore Viol oui elle s'observe du sport amateur jusqu'au plus haut niveau de performance avec dans plus de 80% des cas des victimes mineures, filles et garçons. Et non elle ne sont pas l'exception d'un sport mais un mal transversale à éradiquer dans toutes les disciplines. Si cette lucidité a d'abord demander une prise de conscience collective malheureusement toujours trop lente. Elle a permis depuis d'engager une lutte sans merci pour éradiquer ces violences avec une boussole très Claire qui m'anime chaque jour tolérance 0. Voilà pourquoi ces 3 dernières années nous avons considérablement renforcé notre arsenal d'abord pour ne plus laisser passer ces violences avec la création de la cellule signale sport qui a déjà permis traiter plus de 900 dossiers depuis mars 2020 pour des faits de violence dont 90% à caractère sexuel mais aussi en mobilisant l'ensemble des leviers à notre disposition d'abord judiciaire à travers un signalement systématique au procureur de la République comme l'impose l'article 40 du code de procédure pénale afin que des investigations soient menées, y compris en l'absence de dépôt de plainte administratif ensuite par des inspections et des enquêtes que je n'hésite pas à diligenter à chaque fois puis par des mesures d'interdiction d'exercer ou des fermetures d'établissements sportifs y compris en urgence pour faire cesser les maltraitances et prévenir tout risque de réitération disciplinaire enfin en nous assurant que toutes les fédérations prennent à bras-le-corps leurs obligations de lutte contre ces violences, notamment celles qui ont failli en la matière parfois dans un passé pas si lointain. Notre action collective, soulignons-le, commence à porter ses fruits. D'abord auprès des victimes. Grâce à l'allongement des délais de prescription en 2018 puis en 2021, mais aussi des bourreaux à travers les plus de 400, mesure d'interdiction d'exercer déjà prononcée et plus de 1000 personnes mises en cause. Pourtant des faits extrêmement graves sont encore régulièrement révélés autant grâce aux médias qu'au travers des enquêtes que nous enclenchant ce qui signifie que nous pouvons que nous devons faire mieux encore aujourd'hui je veux donc remercier le sénateur Sébastien Pla pour sa proposition de loi qui est fondée sur cette volonté de renforcer encore davantage notre cadre législatif et qui est le fruit, je tiens à le souligner d'un engagement exemplaire et de longue date de sa part pour lutter contre contre ces violences et à travers vous, vous l'avez dit, c'est aussi à Sarah Abitbol que je veux rendre hommage, chacun sait l'impact et même le choc qu'a représenté sa prise de parole pour le monde du sport. Le début d'un véritable MeToo sportif en lui remettant récemment l'Ordre national du Mérite. Je lui ai dit ceci, nous ne lâcherons rien notamment pour que la libération de la parole s'accompagne ce qui est au moins aussi important d'une vraie libération, de l'écoute. Je tiens aussi à saluer le travail conduit par le rapporteur. Jean-Jacques Lozach, dont je sais l'expertise et l'engagement remarquables sur les politiques publiques du sport, notamment quand il s'agit du respect de l'éthique et de l'intégrité et plus largement l'esprit constructif qui a prévalu dans le cadre de la rédaction de cette proposition de loi car pour lutter contre ces violences. Je suis persuadé que le renforcement du volet répressif doit son compagnon de la plus haute exigence sur le volet également préventif même si chacun le sait le risque 0 n'existe pas d'autant plus qu'un casier judiciaire vierge n'empêche pas de commettre parfois des actes terribles en la matière, ces dernières années, nous sommes déjà monté en puissance en renforçant nos exigences et nos moyens notamment au travers du contrôle d'honorabilité, c'est-à-dire la vérification des antécédents judiciaires visant à s'assurer qu'une personne ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale incapacitantes prévu par la loi et non respectés. Ce contrôle était auparavant limitée aux 250.000 éducateurs titulaires d'une carte professionnelle et suite à la loi du 21 août 2021 confortant les principes de la République, il concerne désormais 2 millions de personnes dont les éducateurs bénévoles dont les juges et arbitres dont les maîtres nageurs titulaire du BNS SA ainsi que tous les intervenants auprès de mineurs depuis près d'un an mais services se sont fortement investis aux côtés des fédérations pour traduire concrètement cette mesure et cette extension sur le terrain nous avons déployé un dispositif efficace largement automatisés qui repose sur la remontée des données d'identité par les clubs et sur un système d'un d'information dédié relatif à l'honorabilité développé par mon ministère en complément les services de l'État réalise régulièrement des contrôles ponctuels sans jamais, je tiens à le signaler pénaliser l'engouement pour le bénévolat sportif ni faire peser sur les clubs locaux de trop fortes exigences. Là encore, les résultats sont là, les 40.000 nouvelle carte professionnelle délivrée en moyenne chaque année aux éducateurs sportifs font désormais l'objet d'un contrôle systématique et s'agissant des bénévoles, les fédérations qui sont très attendus se mettent en ordre de marche, comme en témoigne la multiplication par plus de deux depuis depuis un moment des contrôles réalisés par exemple par la Fédération française de football de boxe ou de Handball au total au 31 mai 2023. Ce sont ainsi près d'un million de personnes qui ont d'ores et déjà été contrôlé et plus de 130 incapacité et mesures de police administrative qui qui ont été prononcées. Pour autant sur ce volet préventif. Nous disposons encore d'un certain nombre de marge de progression et c'est à mon sens toute la force de ce texte que nous examinons aujourd'hui en séance. Il permet d'identifier ces axes d'amélioration si concret qui médias pour lesquels je salue une fois encore le travail réalisé par le sénateur plat et le rapporteur Lozach notamment pour renforcer encore l'équilibre entre le renforcement du rôle régalien de l'État dans son contrôle des personnes intervenant auprès des pratiquants et la responsabilisation accrue que nous souhaitons assurer des instances sportives elles-mêmes pour signaler l'ensemble des faits de violence. Parmi ces propositions d'amélioration. Il convient à mon sens de signaler la consécration au niveau législatif qu'opère ce texte des modalités concrètes de réalisation du contrôle d'honorabilité qui prend la forme d'une interrogation annuel du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes le Fijais fichier qui relèvent tous de du ministère de la justice. 2ème. Exemple, la possibilité de déclarer l'incapacité, même en cas d'effacement du B2 dès lors que la condamnation concernés figurent elle encore au Fijais. 3ème exemple la possibilité pour le préfet d'interdire l'exercice des responsables de APS et non plus seulement de toutes les autres catégories d'acteurs intervenant dans ces établissements ce qui vient combler opportunément un vide juridique. 4ème exemple l'instauration surtout d'une obligation de signalement à l'autorité administrative en cas de comportement d'un encadrant ou de toute personne intervenant auprès de mineurs présentant un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Ce qui est peut être l'apport majeur de ce texte. Cela va permette de systématiser les remontées de faits inquiétants et ainsi pour le préfet de prendre chaque fois que c'est nécessaire, des mesures administratives d'interdiction d'exercer. Enfin monsieur le rapporteur. Vous allez proposer une amélioration par voie d'amendement lors de cette séance publique afin d'intégrer à ce dispositif de signalement une dimension nationale à travers l'obligation pour toutes toutes fédérations agréées de faire remonter les signalements de violences dont elle a connaissance au service du ministère pour en quelque sorte boucler la boucle. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Si le sport est devenu un fait social total pour reprendre les mots de Marcel Mauss, c'est bien sûr du fait des performances des sportives des sportifs mais aussi parce qu'il repose sur des valeurs essentielles, l'émancipation, le respect des règles. Le vivre ensemble. Si nos sportifs travaille dur pour être au meilleur de leur performance. À nous tous de nous mobiliser sans relâche pour être les gardiens du temple de ses valeurs, à un moment en plus critique de l'agenda sportif de notre pays pour avancer sur cette meilleure protection de nos pratiquants. J'ai en effet demandé à Marie-George Buffet, Stéphane Diagana, d'intégrer pleinement cette dimension dans les travaux du comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport qu'il copréside à ma demande et voilà pourquoi enfin dès aujourd'hui. Je me réjouis du renforcement du dispositif global proposé par cette PPL dont je souhaite qu'elle puisse aboutir rapidement à l'Assemblée nationale et je serai extrêmement attentive à la bonne application par l'ensemble des services de l'État et du mouvement sportif de ces dispositions clés je vous remercier. Merci, madame la Ministre, dans la suite de la discussion générale. La parole est à madame Céline Brulin, pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. L'actualité récente nous montre que les violences sexuelles n'épargne pas le milieu sportif depuis 2020 un tournant dans la lutte contre ces violences, a été opéré par le mouvement sportif lui-même et il convient de continuer à doter le mouvement sportif comme la société toute entière d'outils pour lutter toujours plus efficacement contre ces phénomènes. Je veux d'abord saluer celles et ceux qui ont pris la parole pour dénoncer publiquement ce dont ils ont été victimes. On le sait, c'est très difficile mais il faut malheureusement souvent le retentissement de certaines affaires et j'y mets des guillemets pour créer des prises de conscience qui doivent être suivis d'actes forts. La cellule de signalement des violences et des violences sexuelles, créée par votre prédécesseur, madame la ministre a ainsi permis de recueillir 9107 signalements conduisant à 424, interdiction d'exercer. Ça été rappelé vous le poursuivez en créant le comité pour l'éthique et la vie démocratique dans le sport co-présidée par Marie-George Buffet et Stéphane Diagana. Au-delà des chiffres il y a des femmes, des hommes et dans la très large large majorité des cas, des mineurs, c'est-à-dire des enfants et des jeunes venus chercher dans le sport, une source d'épanouissement. Ce que le sport ne devrait jamais cesser d'être. Cette proposition de loi les améliorations pertinentes apportées par le rapporteur comme les amendements que nous allons examiner permettront par exemple de donner une base légale à cette cellule signale sport afin de la conforter, il convient aussi d'en renforcer les moyens Madame la Ministre le contrôle systématique d'honorabilité qui s'applique aux encadrants professionnelle sera élargi aux éducateurs bénévoles qui représentent 90% des éducateurs sportifs il prend modèle sur celui qui s'applique dans le secteur social et médico-social et nous considérons que les modifications apportées à la version initiale de la proposition de loi faisant peser la responsabilité du contrôle sur les services de l'État est particulièrement bien venu, notamment parce qu'il est en effet inutile et même contre-productif de faire contrôler le casier judiciaire d'un intervenant par les dirigeants sportifs eux aussi essentiellement bénévoles plus encore dans le contexte de crise du bénévolat que nous connaissons. D'autant que l'application de la loi sécurité globale, dont nous avions souligné combien les conséquences pourraient être redoutables vient aujourd'hui renforcer nos interrogations tout particulièrement celle stipulant que l'agrément en qualité de dirigeant ou d'associer ne peut être délivrée qu'aux demandeurs dans le bulletin numéro 2 du casier du judiciaire est vierge. La nature des infractions visées surpassant largement l'honorabilité sur laquelle nous légiférons aujourd'hui le sport a souvent montré combien il peut être une source de réhabilitation par les valeurs qu'il promeut l'effort qui l'exige et la satisfaction qu'il peut engendrer ne lui retirons pas cette dimension en cela le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles aux violences Fijais nous semble bon outil est-il utile, comme le fait la proposition de loi de le conforter. les clubs, les fédérations et les ligues ont un rôle à jouer dans la lutte contre toutes les violences et particulièrement les violences sexuelles, mais ce rôle doit davantage tendre à favoriser un environnement serein et protecteur à effectuer les signalements nécessaire à accompagner les éventuelles victimes qu'à exercer des contrôles qui incombe au service de l'État et de ce point de vue la formation des dirigeants et des bénévoles sportifs est indispensable à la prévention là encore des moyens doivent être déployés pour soutenir le mouvement sportif dans cet effort. Nous soutenons cette proposition de loi et nous souhaitons qu'elle permette de gagner en efficacité face aux insupportable violence en particulier sexuelle loin de jeter l'opprobre sur les millions d'acteurs qui font vivre avec dévouement, le mouvement sportif. Nous pensons qu'elle les aidera à se protéger et à protéger tous les pratiquants, notamment les enfants, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Monsieur Pierre-Antoine Levi. Pour le groupe Union centriste pour six minutes.

Monsieur le président, madame la Ministre, monsieur le président de la commission de la culture. Cher Laurent. Monsieur le rapporteur. Monsieur l'auteur de la loi chère Sébastien Pla, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition de loi déposée par notre collègue Sébastien Pla que je tiens à remercier pour son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles sur des enfants. Ces actes abominables aux conséquences dévastatrices persiste malheureusement aujourd'hui. Il est donc essentiel d'améliorer et de compléter la législation existante pour intensifier ce combat. Le sport comme nous le savons tous, est un élément fondamental de l'épanouissement et du développement des jeunes. Leur permet de cultiver des valeurs telles que d'esprit d'équipe, la discipline la persévérance et le dépassement de soi. Cependant certains individus mal intentionnés profitent de cette proximité avec les jeunes athlètes pour commettre des actes inqualifiable et abject. En tant que législateurs, il nous dit, il est de notre devoir de prendre des mesures fermes pour éradiquer ce fléau. Dans sa forme actuelle le contrôle exercé par les clubs sportifs et souvent insuffisants les procédures de vérification des antécédents des encadrants peuvent être lacunaires, permettant ainsi à des individus dangereux de se glisser dans des postes à responsabilité. Est donc primordial que l'État joue un rôle actif dans ce processus de contrôle en mettant en place des protocoles clair et rigoureux pour s'assurer de l'honorabilité des adultes intervenant auprès des mineurs dans le sport. Ainsi, toute personne souhaitant travailler avec des mineurs dans le cadre sportif seraient tenus de se soumettre à une vérification approfondie de ces antécédents. Renforçant le contrôle exercé par l'État, nous enverrons un message fort à l'ensemble de la société. La protection des mineurs est une priorité absolue. Nous ne pouvons plus permettre que des individus manettes exploitent leur position d'autorité pour commettre des actes odieux. Les jeunes athlètes doivent pouvoir s'épanouir dans un environnement sain sécurisé bien. Les statistiques sont alarmantes, selon une étude de l'Institut national d'études démographiques. Plus de 15% des adultes déclare avoir subi des violences sexuelles pendant leur enfance. Dans un cas sur de ces violences engendre des épisodes dépressifs, les troupes de l'anxiété phobique qui rendent difficile la libération de la parole. Plus d'un tiers de ses victimes développe aussi des troupes du comportement alimentaire et un quart de ces victimes tentent de mettre fin à leur vie. Des années a pris la ou les agressions une victime sur six souffre encore d'état de stress post-traumatique ou de trous psychosomatiques. Et pour plus de 5% de ses victimes. Le long processus de désocialisation peut aussi conduire à la rue à la prostitution. Les témoignages courageux de personnalités comme Andréa Bescond et Sarah Abitbol et bien d'autres encore ont permis de sensibiliser le grand public cette réalité insoutenable. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à ces violences sexuelles dans le sport. Les chiffres sont alarmants, 610 affaires ont été signalés à la cellule qui traite le problème des violences sexuelles dans le sport. Depuis sa mise en place en 2020 affaires dans lesquelles 84% des victimes sont des mineurs. D'après les données publiées par le ministère des Sports. 73% des dossiers concernent des faits commis au cours des 10 dernières années et sans cette affaire porte sur la seule saison sportive 2022 1021. Au total, 655 personnes sont mises en cause dont 97% d'hommes. Actuellement 449 dossiers sont clos alors que 206 enquêtes sont en cours. La majorité des fédérations sportives sont concernés. La présente, proposition de loi vise à renforcer le dispositif de contrôle de l'honorabilité des adultes intervenant auprès des mineurs dans des établissements sportifs nous devons exiger un double contrôle à la fois de la part des clubs sportifs. Les services de l'État pour nous assurer de la sécurité de nos enfants. Je suis conscient que certains pouvaient évoquer dans des considérations relatives à la protection de la vie privée. Cependant, il est crucial de souligner que la protection des mineurs doit prévaloir sur toute autre considération. s'encadrants sportifs ont une responsabilité particulière vis-à-vis des jeunes dont ils ont la charge. Il est de notre devoir de nous assurer qu'ils soit digne de cette confiance. Cette proposition de loi prévoit notamment la délivrance annuel les bulletins de du casier judiciaire et d'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Elle prévoit également des mesures pour les personnes condamnées par une juridiction étrangère pour une infraction constituant selon la loi française, un Crime ou l'un des délits mentionnés. Dans le cadre des amendements proposés par le rapporteur je souligne sous je souhaite souligner l'importance de l'amendement IV qui donne une base légale à la cellule signale sport mises en place par le ministère, cet amendement vise à assurer une circulation de l'information à tous les niveaux, permettant ainsi aux fédérations d'être informé sans délai lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne dans le métier en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. De plus, amendement cinq permet de sanctionner administrativement, un président de club qui emploie un éducateur sportif, interdit d'exercer par le préfet, parce qu'ils présente un risque pour les pratiquants. C'est une mesure essentielle pour garantir la sécurité de nos jeunes athlètes. Alors, mes chers collègues, vous l'aurez compris, notre groupe Union centriste votera avec conviction. Cette proposition de loi merci sur Sébastien pour l'avoir présenté, j'espère qu'elle pourra prospérer rapidement pour être appliquée, je vous remercie. Merci. Cher collègue, la parole. Est au président Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE pour 4 minutes.

du patinage de Sarah a du rugby de Sébastien Boyer, tout le monde peut un jour y être confronté, phénomène social. Longtemps considéré comme tabou. Il sort aujourd'hui peu à peu d'un sacré des vestiaires. Grâce à une libéralisation de la parole qui doit permettre à la honte de changer de comme. Je rappelle que chaque année, 170.000 mineurs seraient victimes de violences sexuelles, selon la commission indépendante sur l'inceste. Et les violences sexuelles envers les enfants. Le ministre amateurs comme professionnels ne fait pas exception. Et alimente grandement la liste des victimes. Si Hollande de la sacralisation de la personne de l'entraîneur et c'est de la recherche de la performance une omerta. Il y a longtemps régné la proposition de loi que nous débattons aujourd'hui. Doit accélérer. J'ai pris de conscience et contribuer au tournant, s'opérant depuis quelques années dans la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Le sport, le pouvoir d'offrir une cale universel pour l'apprentissage de valeurs telles que la discipline l'inclusion la part fédérale et le respect il contribue au développement des compétences personnelles nécessaires pour le citoyen était responsable. Il ne doit pas être, à l'inverse, le lieu d'expression privilégié. De prédateur sexuel ou sinon si le communiqué font foi. L'auteur. Alors bon, il faut une loi mais aussi le doigt sur une pour le majeur, l'encadrement du sport français repose principalement sur les bénévoles s'il existe une obligation d'honorabilité pour les éducateurs sportifs professionnels comme bénévoles seuls les éducateurs professionnels font l'objet d'un contrôle systématique annuel répondant aux révélations d'affaires de violences sexuelles qui ont mis en évidence la demande des fédérations sportives et les pratiquants. Quant à la nécessité d'un contrôle de l'honorabilité d'éducateurs sportifs et des exploitants d'établissements d'activités sportives et bénévoles. Le groupe RDSE c'est un toujours voulu le relais éclairé des besoins de nos concitoyens se félicite de cette initiative parlementaire, emporté par Jean-Jacques Lozach. Certes le camp législatif s'est dernièrement renforcée avec l'apparition d'une obligation du recueil de identité complète de toute personne susceptible de devenir éducateur sportif ou d'intervenir auprès de mineurs. Parallèlement, l'apparition d'épidémies. Une cellule de signalement de faits de violence ou nous violences sexuelles a permis le contrôle de l'honorabilité et de la moitié des bénévoles placés au contact des mineurs dans le milieu sportif. Néanmoins, cela reste insuffisant. Je rappelle que si éducateur sportif titulaire d'une carte professionnelle font l'objet de contrôles systématiques réalisées annuellement par une consultation automatisé de leur butin, numéro 2 du quasi judiciaire et de leur fille fût Yes les j'indicateurs sportif bénévole. Les arbitres et exploitable. Du temps misant d'activités physiques et sportives ne sont pas légalement soumis à une content le systématique de cette honorabilité. C'est pourquoi. Par la prise en compte dans le champ sportif des améliorations de la protection des mineurs ici alors attaqué cette proposition de loi met enfin un terme à l'anomalie dont souffrent ce milieu qui repose à 90% sur des bénévoles. Nous pouvons ainsi que nous satisfaire de l'inscription dans la loi du principe annualité du contrôle de l'honorabilité pour tous les intervenants à titre rémunéré ou bénévole auprès des mineurs en milieu sportif, de même que le fait qu'une inscription une condamnation of US Fidesz même si celui-ci n'est plus à ceux qui sont

accélérera responsabilisation. De l'ensemble des acteurs du milieu sportif face à ce phénomène. C'est ainsi que, logiquement, le groupe indien se retrouvera bien sûr cette proposition de loi. Merci monsieur le président. La parole est maintenant à monsieur Jacques Grosperrin pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. je voudrais féliciter Sébastien Pla pour sa PPL et puis. Jean-Jacques Lozach, pour la réécriture globale car la vérification de l'honorabilité est un élément éloquent est important. D'ailleurs ça se traduit par celui qui mérite estime et la considération d'autrui. Je suis heureux qu'enfin il y a une prise de conscience peut-être tardive cap combien d'enfants ont pu être abaissée à ce jour il fallait et il faut contrôler tous ces bénévoles. Mais sur le contrôle de l'honorabilité était prérogatives de l'État, l'inscription dans le Champ sportif des mesures du secteur social et médico-social de la production de l'enfant, la protection de l'enfant est une nécessité. Avec l'obligation de signalement par les présidents de clubs ferment les yeux. Les exemples sont nombreux. Les exemples sont nombreux également sur les présidents de clubs qui ont pu aussi abusé un certain moment des enfants. Je voudrais donc sans état d'âme cette PPL mais suffisant pour protéger notre jeunesse ne sportif. La France souffre du syndrome de Vichy. Nous avons confondu la délation qui consiste à dénoncer de manière méprisable et intéressé avec la dénonciation qui consiste à désigner un coupable à une autorité ou à la justice les anglo-saxons n'ont d'ailleurs jamais eu ces difficultés car la dénonciation est obligatoire dès qu'il y a violence sur un mineur. Madame la Ministre, vous êtes la 25ème Ministre en plus de plein exercice, il y a eu des commissaire. Aux sports avec monsieur Herzog, c'était pas l'Everest. Mais c'était un arbre a vous avez été il y a eu des ministres qui ont été sous tutelle. Tutelle du 1er ministre de tutelle, la qualité de la visite du ministre de temps libre au ministre de la santé et ministre de la ville avec le ministre Kader ministre d'éducation nationale. Je n'ai qu'un regret, c'est que le dernier ministère sur le ministre de l'Éducation nationale de Jeunesse et sport n'ait pas pu s'emparer de ce problème-là parce que c'est le problème aussi de la jeunesse. Je comprends que vous soyez Ministre bien sûr de Ministre des Sports et des Jeux olympiques des Jeux paralympiques, mais j'aurais tant souhaité que soyez également ministre et la jeunesse pour pouvoir justement vous emparer de cette difficulté-là. Car si cette PPL est indispensable pour clarifier responsabiliser chacun il faut aller plus loin. Trop de lois tue la loi disait Pompidou, pouvons-nous contrôler tout le monde y y aura-t-il pas des trous dans la raquette. Quid des sports nous pratiqués dans les fédérations officiel. Quid des écoles de dessin de musique de théâtre etc. Il nous faut inverser le mode opératoire. Il existe trop de lois, je le disais, il nous faut agir plutôt sur l'enfant sous sa construction sur son devenir sur ces représentations. L'école est le lieu de sensibilisation de la prévention. J'ai entendu qu'on pouvait faire des cours d'éducation sexuelle. Créer des ambassadeurs parce que les enfants se confie beaucoup plus à leurs camarades qui a un adulte mais il existe au sein de l'Éducation nationale. Ce qu'on appelle le socle commun des compétences, c'est le cycle qui est obligatoire le l'âge de 3 ans à 16 ans dans ce cycle-là qui doit être maîtrisé avant l'âge de 16 ans qui conduit au diplôme national du brevet, il rassemble un ensemble de valeurs d'attitude nécessaires pour réussir sa vie mais aussi plus exactement et plus important, son avenir de futurs citoyens donc saisi c'est l'opportunité et madame la ministre, avec l'éducation nationale

respect des choix personnel est indispensable et surtout responsabilisation individuelle. Les cours d'éducation physique et participe mais pas seulement les cours de mathématiques, les cours des sciences de la vie de la terre et les cours de les cours qu'on rencontre dans le cadre de l'enseignement obligatoire. Donc il faudra plutôt rédigé et ça ce ne serait peut être de l'ordre réglementaire à une 9e pilier. Soit l'apprentissage de l'appartenance de son corps sur le fait de sa liberté. L'école doit rester un lieu d'échanges. L'école doit être un lieu de libération de la parole parce que je m'interroge. Nous sommes sur une proposition de loi, mais nous pouvons passer sur d'autres propositions de loi, moi je suis judoka alors sur la douleur sur sur les chutes sur les étranglements sur les clés de bras et caetera, sur la souffrance dans le sport. Faisons attention de ne pas légiférer toujours toujours et toujours plus pour poser tellement de problèmes au sport, qui est quelque chose qui est tellement important à nos yeux et que nous espérons que vous serez la ministre non pas des années 1960 avec Rome, où il y a eu aucune médaille d'or, mais où il y aura beaucoup de médailles d'or, merci. Bien en espérant. Monsieur Jacques Grosperrin que personne ne sera étranglée dans cet hémicycle. Je précise qu'un accord avec le groupe socialiste, nous irons au terme de du vote de cette proposition de loi même si nous dépassons évidemment les 13h. La parole est maintenant à monsieur Jean-Pierre Grand. Pour le groupe les indépendants pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, la pratique d'un sport est fondamentale pour l'épanouissement des enfants c'est l'école des valeurs de la vie. Néanmoins, le sport peut engendrer des situations à risques et constituent un terreau favorable à l'apparition de violences sexuelles sur des mineurs, notamment en raison du contexte d'emprise des entraîneurs sur les enfants. Les chiffres sont malheureusement là pour nous le rappeler. Un sportif sur 10 assurent avoir été victime d'agression sexuelle durant sa carrière. Depuis plusieurs années la question des violences sexuelles sur mineurs fait l'objet de travaux par le Sénat qui se monte ainsi. À l'avant-garde et je m'en réjouis. En 2019, la mission commune d'information sénatoriale menée par notre collègue de de Roche avait déjà permis mis en avant la nécessité de renforcer le contrôle de l'honorabilité des adultes en contact avec les enfants. Par ailleurs, en 2021, la loi confortant le respect des principes de la République a instauré un contrôle hein je vois républicain pour les associations, confortant ainsi l'obligation d'honorabilité dans le milieu sportif. Notre devoir en tant que législateur, est de veiller à ce que plus aucun intervenant en milieu sportif placés au contact des mineurs au contact des mineurs n'ait fait l'objet d'une inscription contraire au contact des enfants ou d'une condamnation qu'il aurait omis de déclarer. Tout, absolument tout doit être mis en oeuvre pour lutter contre ce fléau que sont les violences sexuelles dans le milieu du sport. Ainsi le texte que nous examinons aujourd'hui est le bienvenu car il est essentiel d'améliorer la législation existante pour intensifier ce combat en effet le contrôle exercé par les clubs sportifs et souvent malheureusement insuffisantes. Il est donc primordial que l'État joue un rôle actif dans le processus de contrôle en mettant en place des protocoles clairs pour s'assurer de l'honorabilité les adultes intervenant auprès de mineurs dans le sport. Je salue l'excellent travail effectué en commission qui a conduit à réécrire l'article unique en consolidant le cadre juridique de la proposition de loi et en renforçant le contrôle d'honorabilité. Les éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles. Les modalités de ce contrôle sont alignées sur celles des personnes intervenant preuves des publics fragiles. Je partage également la position de la commission qui a souhaité expliciter l'incapacité d'exercer en raison d'une condamnation par une juridiction étrangère je suis favorable à l'article additionnel après l'article unique qui prévoit la création d'une mesure administrative et d'une sanction pénale pour les dirigeants de clubs dans la conduite serait contraire à l'objectif éthique poursuivi Madame la Ministre, mes chers collègues. Les modifications apportées par la par le rapporteur sont très opportune pour sécuriser et améliorer le dispositif initialement proposé le groupe les indépendants votera cette proposition de loi améliorer, consolider juridiquement par la commission. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Thomas Dossus pour le groupe écologiste pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens d'abord à saluer ce travail crucial dans le contexte actuel de libération de la parole qui percute tous les secteurs et pour ce qui nous concerne aujourd'hui toutes les fédérations sportives. Devant la gravité des faits, le caractère parfois insupportables des témoignages la douleur des victimes souvent très jeune à l'époque des faits, nous sommes parfois frappées d'un état de sidération qui peut nous tétaniser mais le silence qui règne sur ce sujet est vécue souvent comme une violence supplémentaire et constante par les victimes, dont chaque occasion de parler des violences commises contre les enfants et d'utilité le sport peut être un lieu d'emprise d'entraîneur d'encadrants ou de coach au comportement criminel et donc les entraînements peuvent devenir un enfer. Pour les enfants. Depuis la prise de parole de la patineuse Sarah Abitbol, la parole se libère et aucune fédération ne semble épargné notre rôle de législateur et donc d'agir, agir pour que la pratique du sport soit protégés en amont des prédateurs pour protéger les enfants. Il faut donc que la peur change de camp et pour qu'elle change de camp. La transparence sur le parcours des encadrants doit devenir la norme, c'est le but de cette proposition de loi après son passage en commission et grâce au travail de notre rapporteur Jean-Jacques Lozach. Le texte nous propose un panel de mesures concrètes pour contrôler l'honorabilité des acteurs du sport car il s'agit bel et bien de contrôler en amont. Ici, l'interdiction pour certaines personnes condamnées. De travailler auprès des enfants dans le sport est en effet déjà codifié au sein de l'article 212 tiré 9 du code du sport aujourd'hui. Il s'agit de le faire respecter. Pour ce faire, il est prévu, le contrôle par l'administration du bulletin numéro 2 du casier judiciaire qui contient la plupart des condamnations judiciaires et des sanctions administratives. Il est également prévu d'appliquer l'incapacité en cas de condamnation à l'étranger, d'ouvrir la possibilité d'une procédure de relèvement c'est-à-dire d'effacement des conséquences d'une condamnation sans que celles-ci ne disparaisse toute la précision que toute condamnation définitive figurant dans le fichier judiciaire automatisé. Des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes entraîne l'incapacité d'exercer, même si celle-ci n'est plus mentionnée dans le casier judiciaire. Le texte prévoit également une mesure administrative d'interdiction temporaire ou définitive de diriger un club sportif pour tout dirigeant qui mettrait en danger des enfants couvrirait un de ces encadrant ou manquerait d'informer l'administration sur les comportements problématiques le concernant. Il prévoit également une sanction pénale en cas de manquement ce panel de mesures nous semble important. Et efficace. Il constitue un 1er pas indispensable pour protéger les enfants pratiquant dans tous les clubs. Au delà de cette PPL importante, il nous faudra aller plus loin dans la protection des mineurs. Il ne faudra développer l'accompagnement des clubs pour la prévention des actes de vols et de violences contre les jeunes sportifs et cela passe par la formation. cela ne se fera pas en un jour. À ce titre, il nous faudra donner formé pardon toute la chaîne des fédérations pour que tous les cadres, souvent bénévoles mettent la parole. Les enfants et leur protection au dessus d'éventuels corporatisme corporatisme ce n'est pas spécifique au sport mais cette libération de la parole doit percer une chape de plomb, le plomb qui a trop longtemps pesé sur ce milieu pour que cet accompagnement, cette formation cette libération de la parole ait lieu, il nous faut naturellement des moyens financiers. Je connais votre engagement Madame la Ministre vous l'avez rappelé, mais je profite donc de cette tribune pour vous appeler madame la ministre, à ce que le prochain projet de loi de finances Bruno connotation significative des budgets dédiés en vous inspirant peut être de ce qu'a fait oh précise au précédent projet de loi de finances. Votre collègue ministre de l'enseignement supérieur de la recherche en doublant les crédits de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce ne sera certainement pas suffisant mais cela permettrait d'enclencher dans les faits dans les projets un palier. Dans la lutte contre ces violences en définitive nous voterons pour la présidente précise, proposition de loi dans sa version réécrite par les amendements du rapporteur. Celle-ci est une première étape indispensable avant d'aller plus loin pour pour la suite, je vous remercie. Merci. Cher collègue, la parole est maintenant Madame Samantha Cazebonne pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. En 2022 60 % des Français de 15 ans et plus. Pratiquer une activité physique et sportive régulière en 2018 40 % des pratiquants sportifs étaient des enfants. La pratique d'un sport est fondamental pour le développement des enfants bien évidemment d'un point de vue de santé mais également en tant que vecteur de lien social, de vivre ensemble et d'épanouissement. En Europe, près d'un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles. Le monde du sport n'est malheureusement pas en reste et près d'un sportif sur 10 déclarent avoir subi des violences sexuelles. L'enfance a été placé par le président de la République au nombre de priorités du nouveau quinquennat et la protection des droits des enfants est au coeur de la feuille de route du gouvernement qui en fait un engagement fort est prioritaire par ailleurs, je tiens à souligner l'engagement du ministère des sports qui a fait de la lutte contre les violences sexuelles, une priorité de son action. En janvier 2020, Sarah Abitbol championne de patinage artistique dénonce dans son livre un si long silence avoir été violées agressées et harcelées par son ex-entraîneur. Cette prise de parole a déclenché le MeToo, du sport et une cellule a été créée par le ministère des Sports en février 2020 afin de recueillir la parole de victimes de violence dans le sport. 3 ans après l'ouverture de cette cellule près de 1000 signalements de violences sexuelles dans le sport ont été effectuées selon les travaux de la commission de lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans le sport, créé par le comité national olympique. Néanmoins, selon la co-, présidente de cette commission. Il faudrait multiplier le chiffre par 10. Pour être fidèle à la réalité. En effet, tous les chiffres et statistiques sur les violences sexuelles sont à prendre avec beaucoup de précaution, compte tenu de la difficulté pour certaines victimes de relever. De révéler pardon ce qu'elles ont subi la libération de la parole des violences sexuelles dans le sport a été suivi de la mise en place de dispositifs permettant de lutter contre ce fléau ainsi plusieurs arrêtés sont venus renforcer le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs et exploitants d'établissements d'activités sportives. Physiques et sportives bénévoles, via notamment le système d'information automatisés du contrôle d'honorabilité. Néanmoins, jusqu'à présent, seuls les éducateurs professionnels faisait l'objet d'un contrôle systématique annuel Le sport français repose à 90% environ sur des et d'éducateurs sportifs bénévoles. Ainsi l'objectif de cette PPL. De s'assurer que tous les éducateurs et intervenant en milieu sportif bénévole où professionel placé au contact des mineurs ne font pas l'objet d'une inscription au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violence ou d'une condamnation qui leur interdit d'y exercer les travaux de la commission que nous saluons ont ajouté une obligation pour les dirigeants de clubs sportifs, à signaler tout comportement à risque des bénévoles employer des mesures administratives d'interdiction exercer pour tout dirigeant de club qui exploiterait un éducateur sportif au mépris du contrôle d'honorabilité refuserait de signaler des comportements à risque dans son club ou qui présenterait lui-même un danger pour la sécurité et la santé morale et physique des pratiquants. Par ailleurs, la commission a laissé à la responsabilité de l'État d'effectuer les contrôles d'honorabilité annuel, estimant que ces contrôles ne pouvait rêver relevait de la prérogative unique des clubs sportifs Le texte que nous examinons aujourd'hui renforcera effectivement la protection des mineurs dans le sport par des contrôles d'honorabilité effectif et annuel afin de protéger les mineurs au mieux dans leur pratique sportive. Le groupe RDPI votera en faveur de ce texte qui prolonge et renforce l'indispensable combat contre les violences sexuelles dans le sport. Merci. Si cher collègue. La parole est maintenant à madame Sabine Van pour le groupe socialiste pour six minutes.

Monsieur le Président Madame la Ministre. Monsieur le président de commission messieurs. Les rapporteurs et auteur de cette PPL, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord rendre hommage à l'auteur de cette proposition de loi notre collègue Sébastien Pla. Il a travaillé avec l'ex-sportif de haut niveau et patineuse artistique, Sarah Abitbol qui, en 2020. A dénoncé les viols qu'elle a subi de la part de son entraîneur d'autres courageuses athlètes isolé comme la tennis woman Isabelle Demongeot le rugbyman Sébastien Boueilh là. L'athlète Emma Oudiou ont permis grâce à leur révélation que se brise la loi du silence qui régnait dans le monde du sport. Il était en effet particulièrement difficile pour les jeunes de parler d'actes subis par une personne de confiance et nous savons qu'un enfant sur 7 serait victime de violences dans le monde du sport. Depuis 2020 il y a eu une véritable prise de conscience de la nécessité de lutter contre les violences sexuelles dans le sport avec la création de la cellule de signalement des faits de violence et de violences sexuelles qui a conduit à la fin 2022 à 904 signalements et 424 interdiction d'exercer. Je rappelle que 90% des éducateurs sportifs sont des bénévoles et que jusqu'en 2022. Ceci n'étaient pas contrôlés systématiquement seuls les éducateurs professionnels l'été une fois par an. Ainsi je me félicite qu'à la fin mai 2023 ans plus de 1 million de bénévoles étaient contrôlé. C'est une nouvelle orientation plus que souhaitable et nécessaire. Notre proposition de loi s'inscrit dans ce vaste mouvement de prise de conscience de la nécessité de lutter contre les violences et violences sexuelles dans le sport. Elle entend donc entouré de davantage de garanties le recrutement des personnels enseignants animant et encadrant des activités physiques et sportives en renforçant leur contrôle d'honorabilité. L'objectif de ce texte et d'éviter qu'un seul encadrant sportif ne passe à travers les mailles du filet. Faute de contrôle. Pas assez systématique ou alors incomplet. Cette proposition de loi qui veut renforcer l'éthique dans le sport et particulièrement bienvenu au moment où la France va accueillir la Coupe du monde de rugby puis les Jeux olympiques et paralympiques le dispositif original de notre PPL prévoyait l'obligation pour les dirigeants des clubs de sport de procéder à un contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs et des intervenants auprès des mineurs. Avec la présentation du bulletin numéro 3 du casier judiciaire avant toute prise de fonction, il appartenait aux dirigeants sportif de vérifier l'absence de condamnation, entraînant une incapacité d'exercer sous l'impulsion de notre rapporteur Jean-Jacques Lozach, dont je salue la qualité du rapport. Nous avons adopté en commission son amendement de réécriture du dispositif de la PPL ainsi le contrôle de l'honorabilité demeure une prérogative de l'État. Cette lourde responsabilité ne devant pas peser sur les épaules de dirigeant sportif très souvent bénévoles le contrôle du bulletin judiciaire trois par les dirigeants de clubs et donc supprimer d'autant que sa consultation ne garantit pas l'honorabilité du futur éducateur sportif cette réécriture à aligner les modalités de contrôle des éducateurs sportifs sur celle applicable au secteur médico-social, ainsi l'inscription d'une condamnation au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes le Fijais entraîne une interdiction d'exercer. Même si cette condamnation ne figure pas sur le bulletin judiciaire numéro deux, dont certaines condamnations peuvent d'ailleurs être effacées au bout de 6 mois cette réécriture renforce incontestablement la protection des mineurs tout comme la nouvelle disposition introduite sur l'interdiction d'exercer lorsqu'il y a une condamnation à l'étranger pour des faits qui en France entraîne la capacité d'exercer l'amélioration du dispositif de lutte contre les violences sexuelles se confirme encore avec l'adoption en commission d'un autre amendement de notre rapporteur créant un article additionnel à cette PPL cet article, introduit une mesure administrative d'interdiction temporaire ou définitive de diriger un club lorsque le comportement du dirigeant est à risque pour les pratiquants lorsque celui-ci maintien dans l'emploi, un éducateur ne respectant pas les critères d'honorabilité ou ne signale pas à l'État un éducateur sportif ou un intervenant présentant un danger pour les jeunes pratiquants. Actuellement, les préfets peuvent seulement fermé administrativement les clubs mais rien n'empêche les dirigeants d'ouvrir un autre club. Je me félicite de ces améliorations voté à l'unanimité en commission qui illustre notre volonté commune d'être à l'écoute de l'ensemble des acteurs, tous mobilisés pour lutter contre ces fléaux des violences et violences sexuelles dans le sport avec des solutions concrètes au plus près du terrain. Je serai attentive à madame la ministre, dans le cas des prochaines discussions budgétaires à votre engagement de doubler les effectifs dédiés de votre ministère pour assurer le contrôle d'honorabilité. Notre groupe votera cette proposition de loi améliorer, consolider juridiquement par notre travail. Pragmatique commun. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Michel Savin. Pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre, Monsieur le Président de commission. Monsieur le rapporteur, maire, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui donc une proposition de loi de notre collègue socialiste Sébastien Pla. Proposition de loi sur laquelle toutes les tendances politiques pourront se retrouver puisqu'il s'agit de renforcer la protection des mineurs. Ici, dans le cas des activités physiques et sportives. Le Parlement réaffirme à cette occasion son soutien plein et entier aux victimes de violences sexuelles à ses victimes. Nous disons qu'elles ne sont ni responsables ni coupables. C'est pourquoi il est de notre rôle de traduire ce soutien dans la loi à chaque fois que nous le pouvons, en facilitant le signalement en punissant plus durement les auteurs de violences en consolidant la prévention et en permettant aux acteurs de terrain d'agir. Le plus tôt possible la libération de la parole a été une une onde de choc a débouché sur une prise de conscience irréversible ce mouvement a ouvert les yeux a beaucoup et d'a surtout permis aux victimes de mettre des mots sur leur expérience et sur leur douleur. De nombreux sportifs et sportifs ont pris la parole pour témoigner de faits d'agressions sexuelles à des époques différentes d'indiscipline très éloignées et avec à chaque fois des mécanismes de domination et des spirale de violence qu'on retrouve très trop souvent. Du chemin reste à parcourir. C'est vrai mais le Sénat avance avec des détermination sur ce chemin vers plus de justice et de sécurité de tous. Armés 2019 une mission d'information sénatoriale présidée par notre collègue Catherine Deroche avait proposé 38 propositions pour mieux protéger les enfants contre le risque d'agression par des adultes dans le cadre de leur métier. Au-delà de la sensibilisation effectué auprès des mineurs et de leurs parents, de la formation des encadrants, l'un des principaux leviers pour protéger les jeunes pratiquants et le contrôle d'honorabilité des personnes qui les entourent. Dans le cas des activités sportives auxquelles il participe. Cette proposition de loi bien donc éteindre ce contrôle automatisé de l'honorabilité des licenciés exerçant dans des fonctions d'éducateur sportif à tous les adultes encadrants ou non qui sont au contact des mineurs au sein des établissements dans les caisses sont pratiquer des activités physiques aux sportive par ailleurs ce texte oblige les présidents de club signaler aux services de l'État, les comportements d'éducateurs de bénévoles de licencier, qui pourrait présenter un danger pour les mineurs. Enfin, cette proposition de loi crée une mesure administrative d'interdiction. Temporaire ou définitive d'exercer pour un dirigeant de club qui passeraient outre les obligations des vérifications d'honorabilité pour l'emploi de ces éducateurs sportifs. L'idée étant de sanctionner ceux qui ne respecteraient pas ce contrôle d'honorabilité qui mettraient leur licenciés mineur en danger. Cette mesure permet également d'éviter toute fermeture administrative de clubs et devrait d'autre part sécuriser juridiquement le représentant de l'État dans sa prise de décisions d'interdiction d'exercer. Je souhaite saluer la réécriture de cette proposition de loi en commission par notre rapporteur dans sa version initiale, ce texte faisait peser un trop important sur les dirigeants de clubs et les fédérations en leur imposant de demander un bulletin numéro 3 du casier judiciaire aux éducateurs et bénévoles intervenant auprès des mineurs. Il s'agissait d'une responsabilité supplémentaire pour les responsables de clubs sportifs qui comptent dans leurs rangs un grand nombre de bénévoles faisant vivre leur leur club partout sur le territoire comme nous l'avons évoqué en commission ce poids supplémentaire présenter un risque à terme pour la survie des clubs qui peinent à trouver des personnes pour les animer reste en suspens, madame la Ministre, sur la question des bénévoles non licenciés dans les dans les clubs et qui interviennent de façon régulière ou partiel. Auprès des enfants et qui peuvent passer au travers encore du mailles du filet. Dernier point, je souhaite a-t-il personnel exprimer mon désaccord en ce qui concerne un amendement que nous allons étudier dans quelques minutes. En effet, je ne suis pas favorable à cet amendement qui prévoit d'exclure de la liste des infractions fixées par l'article 1 de l'article L 212 tiré 9 du code du sport. Une personne qui a participé à un attroupement après sommation et qui a fait l'objet d'une condamnation au vu du code pénal qui prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, après être passé devant un juge qui a pris sa décision sur la base des faits sur ce point je souhaiterais avoir l'avis du du gouvernement sur cet amendement, pour conclure avec mes collègues du groupe LR nous partageons donc les ambitions de ses textes et saisissons cette opportunité qui nous est donné pour protéger les plus fragiles et si plus particulièrement les mineurs. C'est pourquoi nous voterons en faveur de ce texte. Merci, chers collègues, la discussion générale est Close. Nous passons au texte de la commission et à l'article premier je suis saisi d'une demande de parole du président Jean-Claude Requier. Ah si monsieur le président. Ma, mes chers collègues, cette rubrique de par le monde Nathalie Delattre chaque année ce sont plus de 50.000 personnes, le plus souvent jeunes qui se forment au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur le Barça ou au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur le BAFD ces diplômes sont dans une certaine mesure indispensable pour pouvoir intervenir dans les accueils collectifs de mineurs en effet

doivent respecter un cahier des charges comme bon comprendre. Critères où figure notamment la formalisation d'un projet éducatif qui promeut la liberté de conscience et la non-discrimination, or ce sont chaque année plusieurs centaines de mineurs qui sont victimes d'agressions sexuelles de la part des ânes qui Abraham titulaires ou stagiaires dame Barbara ou dans ce milieu où on ne Martin reste très présente la hiérarchie. Ou. Bien trop souvent de la politique de l'autruche. Face à ce constat, alors ai dit c'est des critères sont codifié à l'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 2015 relatives au brevet d'aptitude fonctionne. De directeur un accueil collectif de mineurs Nathalie Delattre appelle le gouvernement à porter attention à cette problématique et compléter cette liste fait de conditionner l'habilitation délivrée à un 2ème critère relatif à la formation des futurs animateurs et directeurs à un plan de prévention des violences sexuelles.

monsieur Sama. On a déjà parlé mais je vais descendre cet amendement. Je l'ai dit en en discussion générale la présente, proposition de loi vise bien au contrôle de habilité plus que l'honorabilité elles-mêmes. En effet, selon l'article 210 12 tiré 9 du code du sport. Il est déjà interdit de travailler dans le monde du sport auprès des enfants, personnes condamnées pour une liste longue d'infraction, la plupart n'appelle pas de commentaire particulier car ce sont des crimes et délits très graves. En revanche, lorsqu'on regarde en détail notamment dans le livre IV du code pénal, il y a là des infractions qui nous semble assez éloigné de l'objectif initial du titre de cette proposition de loi, la protection des mineurs, notamment le fait de participer à un attroupement après sommation. Et donc, je sais bien que la liste de l'infraction n'est ni le fait de l'auteur de la proposition de loi ni du rapporteur elle peut exister à la PPL au sein de l'article du Code du sport que j'ai cité et donc on nous souhaitons symboliquement au moins retiré le fait de participer à un attroupement après sommation de la liste de des des des infractions. Merci. Avis de la commission. Monsieur le rapporteur. la ville de la commission et est favorable JB. Les les arguments de notre collègue Michel Savin. Mais je tiens à apporter de deux 3 précisions donc cet amendement il vise à exclure de la liste des délits écrivent entraînant une incapacité exercer la fonction d'éducateur sportif le fait lors d'une manifestation de ne pas se disperser, malgré les sommations de le faire. Je tiens à préciser que cela ne concerne que des personnes non armées l'amendement vise seulement l'article 431 tiré 9 du code pénal. Le fait de participer armée à une manifestation continue d'entraîner une incapacité d'exercer la fonction d'éducateur sportif, ce délit d'ailleurs défini à l'article 431 tiré 10 du code pénal. Par ailleurs, il existe un délit spécifique à la dissimulation volontaire du visage au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risque d'être commis. Cette disposition a été introduite par la proposition de loi de notre collègue Bruno Retailleau sur le maintien de l'ordre lors des manifestations de 2019. Ce texte, ça crée un nouveau délit de dissimulation volontaire du visage à l'article 431 9 1 du code pénal qui figure toujours parmi la liste des articles du code pénal, entraînant une incapacité d'exercer cet amendement ne vise donc pas à permettre à des Black blocs de devenir éducateur sportif il prend seulement en compte le fait que des enfin une manifestation sont parfois chaotique et que des manifestations des manifestants pas toujours à se disperser malgré les sommations. Donc voilà un peu le, le sens de notre avis favorable en commission. Merci. Avis du gouvernement. Madame la Ministre. Monsieur le président, Monsieur le le sénateur. Avis défavorable. En ce qui nous concerne, pourquoi vous proposez de supprimer l'infraction de participation à un attroupement après sommation. Au motif. Que cette infraction n'aurait aucun lien avec la protection des enfants. Face à ces problématiques de violences sexuelles dans le sport. Mais en réalité le dispositif. Prévu par le code du sport et que nous revoyons aujourd'hui ne vise pas uniquement à protéger les enfants. Mais bien l'ensemble des pratiquants et ceux-là, face à toutes les formes de violence. Le titre de cette PPL c'est la protection des mineurs mais aussi et le contrôle de l'honorabilité. N'ouvrons pas là un espace une brèche là où on a essayé sur le reste du texte de les refermer le plus possible Que l'infraction que vous souhaitez exclure. Elle est vraiment loin d'être anodine. Il s'agit de. Un attroupement illégal après plusieurs sommations par les forces de l'ordre. C'est une incivilité grave qui est contraire aux lois de la République qui est source de trouble à l'ordre public, raison pour laquelle d'ailleurs, ce délit est puni d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende. Dès lors, il me paraît très sincèrement nécessaire que ce délit soit maintenu dans la liste des condamnations incapacitantes bien sûr dans notre ordre républicain, sous le contrôle du juge judiciaire qui peut toujours appréciée souverainement. Les faits pour le cas échéant écartés ou pas les auteurs de tels faits de mission en lien avec le service public dans le Champ sportif. Je pense qu'il faut qu'on soit cohérent jusqu'au bout.

Notre volonté. Moi volonté mais c'est vrai que je pense que le groupe va. Le suivre ça pas d'exclure. Des personnes qui vont manifester et qui. Peuvent arriver à se retrouver. Du fait de la fin d'une manifestation. Avec d'un côté des forces de l'or, de l'autre côté des manifestants. Et puis qui sont. Récupérées pas la police ou la gendarmerie mais qui sont pas condamnées, ces gens-là ne sont pas touchés par le texte. Ceux qui sont touchés par le texte et ceux qui sont condamnés par un délit moi je pense qu'il ne faut pas ouvrir cette porte parce que comme vient de l'oral c'est pour ça que je remercie Madame la Ministre de de de donner votre position parce que si on commence ouvrira la porte à ceux qui. Lors d'une manifestation sont condamnés qui se passe devant un juge, le juge juge. Décide de condamner cette personne avec un an de prison et 15.000 euros d'amende, c'est qu'il y a eu des faits graves, soit d'agressions soit de casse et aux deux donc on ne peut pas confier.

des fois ça parfois récupéré pas les polices mais qui sont libérés rapidement c'est pas cela, donc c'est bien ce qui sont jugés et condamnés. Donc je je souhaite moi que cet amendement soit rejeté pour qu'on évite toute. Ambiguïté sur ce type de comportement. Merci président. Moi j'ai repris le dictionnaire et sur la définition de l'honorabilité, c'est qui mérite l'estime et la considération d'autrui. Moi je m'interroge et ce qui a véritablement estime et considération d'autrui dans la mesure où

ou de 15.000 euros d'amende. Je crois qu'il y a une valeur idiote. En tout cas il y a un exemple donné il y a la valeur de l'exemple pour un éducateur comme un éducateur peut partir avec un masque avec une avec un emprisonnement ou avec une en tout cas une punition quelque part et revenir de manière très simple, faire cours avec des élèves, ça dénote, en tout cas. Certaine perception de la personnalité. Alors chacun a le droit de faire ce qu'il veut mais je pense que la valeur d'exemple doit primer dans le sport et on en parle souvent. Chez les enseignants, il y a certes un engagement de déontologie, je pense chez les éducateurs aussi il doit y avoir un enseignement en tout cas une notion de de de déontologie pardon à respecter et c'est pour ça que je pense je pense qu'il faut voter contre cet amendement. Monsieur Lévy. Oui, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues, effectivement, au vu des explications données par Madame la Ministre. Sur les conséquences qui pourraient arriver avec la le vote de cet amendement. Les explications de Michel Savin. L'idée n'est pas et je trouve le. La présentation de notre rapporteur extrêmement louable puisqu'elle visait à exclure sur. Sur des films considérés comme étant pas grave mais là on est effectivement dans la notion de condamnation notion de condamnation. Attroupement et après sommation. Effectivement, Madame la Ministre, mes chers collègues, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une exemplarité totale quand on est encadrant et donc effectivement, au vu de ces éléments au vu de ce changement. De paradigme. Je pense qu'il nous faut rejeter cet amendement. En tout cas, nous voterons contre. Madame brûle hein. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je pense que nous devrions tous faire preuve d'un peu de discernement. Je rejoins complètement les arguments développés par le rapporteur. Il ne s'agit évidemment pas de faire en sorte que des Black blocs encadre demain. Des jeunes dans nos clubs sportifs mais nous avons tous des témoignages. Nous avons même pour certains d'entre nous parfois vécu. Le fait de se retrouver dans des manifestations qui se termine. À notre corps défendant, pas toujours très bien. Et de se retrouver un peu piégé dans certaines situations, vous avez peut-être lu comme moi le témoignage d'une jeune femme qui en sortant d'une séance de sport s'est trouvé je précisément dans une manifestation plus ou moins organisés, j'en conviens. Et qui c'est qui a eu maille à partir avec la justice pour cette raison-là, alors qu'elle se trouvait là totalement par hasard. Et donc je pense qu'il faut faire attention à ça, enfin moi j'ai en commission, j'ai interrogé sur le terme d'honorabilité. Depuis on m'a expliqué que c'était le terme juridique il convenait. Pour les sujets que nous traitons aujourd'hui mais. La définition que vient d'en donner. Jacques Grosperrin ne me semble pas être la bonne parce que. Lequel d'entre nous est habilitée à juger de l'honorabilité dans les termes qu'il a évoqué de telle ou telle pour encadrer. Des jeunes dans des clubs sportifs et donc oui absolument oui a empêché. Des prédateurs. D'encadrer des enfants de comme nous l'avons tous dit d'être. Sans concession. de de travailler utilement pour protéger les sportifs en général les enfants et les jeunes en particulier mais avec discernement ne rajoutons pas. Du chaos au chaos. Merci je suis saisi d'une demande de scrutin public sur cet amendement numéro 1 Madame la Ministre vous vouliez vous exprimer. je souhaitais re-indiqué que on parle bien d'une condamnation. Ce qui veut dire que la personne en question a été interpellé, qu'elle a fait l'objet d'une enquête que son intentionnalité a été établi et que sa culpabilité a été a été établi, encore une fois on ne parle pas d'un simple militant manifestant pour une cause. Elle est exceptionnellement monsieur Dossus une fois que normalement le scrutin est appelé. Oui, s'exprime plus mais alors. Mais en fait le, ce que ce que ce que ce qu'a dit Madame. Il suscite un commentaire. Il suffit d'avoir lu des comptes rendus ou d'avoir assisté à des comparutions immédiates. Après un certain nombre de manifestations qui se sont mal terminées pour comprendre que les jugements dans c'est sur circonstances là sont parfois des jugements. À la volée et pas forcément très représentatif du droit et de l'enquête que vous appelez de dans dans votre commentaire. Donc et et encore une fois un certain nombre de délits et ont été. Amalgamé à à ma proposition et effectivement c'est pas c'est c'est c'est pas très sérieux. La façon dont, dont ça a été présenté, mais bon, je prends acte. Maintenant de du vote en cours. Très bien donc je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. Le scrutin est ouvert. Appel qui a un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement.

Ça ne demande à voter. Le scrutin est clos. Sur cet amendement votants 343 exprimés, 333 pour l'amendement 92 contre 241. L'amendement n'est pas adopté. Je mets maintenant aux voix l'article 1er de cette proposition de loi qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté à l'article de un amendement IV de la Commission monsieur Oui, monsieur le président. C'est donc un, un amendement qui donne tout simplement une base légale à la cellule signal sport qui a été mis en oeuvre par. Le ministère ces dernières années et on l'a rappelé, dans nos interventions liminaires réciproque. Elle a véritablement fait fait ses preuves et puis d'autre part, cet amendement. Inclut une obligation de signalement de de la part des fédérations et vise à mieux faire circuler l'information entre les différents niveaux. Merci avait. Du gouvernement Madame la ministre. Qui suis favorable et je remercie le rapporteur pour cette proposition. Je mais aux voix l'amendement IV de la Commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté un amendement cinq également de la commission. Monsieur le rapporteur. De la sanction administrative du, du président du club. Un président qui emploie réelle d'éducateur sportif interdit d'exercer par le préfet donc par l'autorité administrative parce qu'il présente un risque pour les pratiquants. Donc il s'agit là de de compléter tout simplement la sanction administrative que nous avons créée par la commission. Merci avait du gouvernement Madame la ministre. Avis favorable. J'ai même indiqué dans mon intervention d'ouverture que c'était pour moi l'un des traits majeurs. De ce texte. Je mais aux voix l'amendement. De la Commission avec un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 2 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je suis saisi d'une demande de scrutin public. À la demande du groupe socialiste. Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Votants 343 exprimés, 343 pour 343 contre 0. Le texte est adopté à l'unanimité. Oui

Écoutez c'est c'est un match que nous avons joué en équipe avec engagement est clair et respect surtout ça donne une très belle image du sport. Ce que nous venons de de vivres ce maintenant donc c'est un pas de plus dans la lutte contre les violences sexuelles. Sur mineurs et sur la question du contrôle d'honorabilité, c'est, c'est un geste fort un soutien aux victimes et aux associations de victimes puisque nous sommes là aujourd'hui, c'est, c'est aussi parce que eux ont le courage de parler. Et puis c'est aussi, il y a c'est un signal très fort en direction des prédateurs sexuels pour qu'ils sachent que les pouvoirs publics.

Dans le monde sportif. Je voulais remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à ce sujet au courage des victimes au ministère pour. Les échanges que nous avons eu dans la co-construction du de ce projet à mon groupe politique d'avoir. Décidé de de choisir de sélectionner notre notre PPL dans notre niche parlementaire au sénatrice Au et o l'ensemble des sénateurs de la commission culture belle commission Culture et éducation pour pour ses apports à Agen Jacques mon ami Jean-Jack et ses équipes pour pour son travail. Une pensée à à en direction de Pauline administratrice qui a fait un travail remarquable avec nous nous accompagner. Une pensée aussi à à mes équipes Alain samedi les petits puis ça fait 2 ans et demi que nous travaillons sur ce sujet et puis enfin à Sarah, Sarah Abitbol que je tenais à excuser qui m'a demandé de l'excuser parce qu'elle elle vient de finir sa, c'est sa tournée. Holiday on Ice et elle prendre du repos. Aux États-Unis, à Miami. Je ne doute pas que depuis bas elle elle doit être très très très heureuse de l'encouragement que ce que le vote unanime de ce texte a fait l'objet aujourd'hui vraiment merci du fond du coeur à toutes et à tous merci beaucoup. Merci cher collègue. Chers collègues Madame la Ministre je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h 45 pour l'examen de la proposition de loi visant à mettre en place un registre national des cancers en fonction de l'ordre du jour réservé du groupe Union centriste. La séance est suspendue.